La séance est reprise. L'ordre du jour appelle la désignation des membres d'une mission d'information et de deux commissions d'enquête. En application des articles 8 et 8 , alinéa 5, du règlement, les listes des candidats remises par les groupes politiques pour la désignation des membres de la mission d'information sur le thème « Comment redynamiser la culture citoyenne ? de la commission d'enquête sur l'influence croissante des cabinets de conseil privés sur les politiques publiques et de la commission d'enquête « afin de mettre en lumière les processus ayant permis ou pouvant aboutir à une concentration dans les médias en France et d'évaluer l'impact de cette concentration sur la démocratie » ont été publiées. Ces candidatures seront ratifiées, si la présidence ne reçoit pas d'opposition dans le délai d'une heure prévu par notre règlement. En accord avec le groupe Écologiste - Solidarité et Territoires, la désignation des dix-neuf membres de la mission d'information sur le thème « Protéger et accompagner les individus en construisant la sécurité sociale écologique du XXI siècle » aura lieu mardi 23 novembre, à quatorze heures trente, le délai limite pour la remise des listes de candidats étant fixé le même jour, à dix heures. Il n'y a pas d'opposition ... Il en est ainsi décidé. J'informe le Sénat que des candidatures pour siéger au sein de l'éventuelle commission mixte paritaire chargée d'élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2021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

où il est fait référence à votre dernier ouvrage dans lequel vous suggérez, à propos de la réforme des institutions et des pouvoirs du Parlement, de « limiter les compétences du Sénat en matière budgétaire à des observations et à une approbation finale, et non plus une lecture complète »

Madame la présidente, monsieur le président de la commission des finances, monsieur le rapporteur général, monsieur le ministre délégué- je vous propose de laisser à une prochaine séance, qui risque d'être longue et houleuse, la discussion sur l'organisation institutionnelle du pays. Je suis gaulliste, j'ai des convictions gaullistes et, en ce qui concerne la place du Sénat

les résultats économiques de la France. Nos résultats économiques sont là : 6,25 % de croissance prévue pour 2021,

Les investissements des entreprises redémarrent, la consommation est forte. Nous avons donc devant nous une perspective de redressement économique dynamique, avec une France qui tire les autres économies de la zone euro. euro. Ces résultats économiques sont, d'abord, dus au travail de fond que nous avons engagé en début de quinquennat, notamment la baisse des impôts sur les ménages comme sur les entreprises qui incite à consommer et à investir. dus, ensuite, à la vigueur du plan de relance que nous avons mis en place, dont 70 milliards d'euros seront engagés dès la fin de l'année 2021. Ils sont dus, enfin, au plan d'investissement que nous avons commencé à déployer. Il existe néanmoins des risques que je voudrais rappeler à cette tribune. Le premier risque, chacun en a conscience, c'est le retour de la pandémie. Je voudrais une nouvelle fois appeler chacun au sens des responsabilités, à la vaccination, dont le rappel vaccinal, et au respect des gestes barrières pour éviter que nous ayons à revivre en fin d'année 2021 ce que nous avons connu l'année dernière. Je me souviens très bien de ces semaines de l'année dernière, où nous étions tous confrontés à des fermetures de commerces et aux difficultés des artisans, des indépendants, des grands magasins, des grandes surfaces, Je ne voudrais pas qu'à quelques semaines de Noël, alors que tous ces secteurs d'activité redémarrent remarquablement bien, que les restaurants embauchent et cherchent des employés, que les commerces préparent les fêtes de Noël, les fêtes de Noël, la pandémie nous oblige de nouveau à des restrictions qui pèseraient sur la vie de nos compatriotes. Je crois que c'est aujourd'hui le risque principal. Il dépend de chacun d'entre nous et de notre sens des responsabilités. Le deuxième risque qui pèse sur la croissance française, c'est le risque de pénurie de main-d'oeuvre et de composants, notamment de composants électroniques et de semi-conducteurs. vous en êtes tous fait l'écho au cours des dernières semaines. L'ajustement prendra du temps- on ne règle pas les problèmes de main-d'oeuvre du jour au lendemain -, en particulier sur les semi-conducteurs qui sont essentiels pour toute industrie, automobile comme aéronautique. La seule bonne réponse consiste à mener une politique d'investissement de long terme pour que la France puisse disposer des semi-conducteurs dont elle a besoin pour son industrie, ses transports, ses télécommunications. C'est exactement ce que nous avons commencé à engager

Enfin, le troisième risque, celui dont on débat beaucoup, c'est celui de l'inflation. Je veux le confirmer à cette tribune, notre évaluation est que l'inflation est temporaire. est temporaire. Elle est tirée principalement par les prix de l'énergie et, dans le fond, la véritable difficulté est moins la hausse des prix que la forte augmentation des prix spécifiques de l'énergie, qui appelle des réponses fortes et rapides comme celles que le Gouvernement a apportées. Pour le coup, cette augmentation des prix de l'énergie s'inscrit sur plusieurs mois. En effet, la demande est très dynamique en Chine, aux États-Unis et partout en Europe. En outre, l'épuisement des ressources fossiles, les moindres financements en faveur de ces énergies ou encore la transition vers des énergies renouvelables

Par conséquent, il n'y a pas à craindre de contagion automatique de l'augmentation de l'inflation des États-Unis vers l'Union européenne. En somme, mieux vaut une analyse lucide que d'exagérer la gravité de la situation ; mieux vaut garder son sang-froid sur ce sujet très sensible de l'inflation. C'est ce qui nous a amenés à apporter deux réponses spécifiques : l'une sur l'énergie et l'autre en direction des ménages les plus modestes. Sur l'énergie, d'abord, le Premier ministre a annoncé le gel des prix du gaz et le plafonnement des prix de l'électricité, qui est absolument vital, puisque, aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, nous sommes confrontés à une augmentation des prix de l'électricité qui pourrait atteindre plus de 15 % à la fin Nous avons garanti aux Français que l'électricité n'augmenterait pas de plus de 4 % à cette échéance : nous prendrons à notre charge la différence entre ces 4 % et l'augmentation automatique. Je veux insister aussi, toujours sur la réponse à apporter en matière d'énergie, sur la nécessité de modifier en profondeur le marché européen de l'énergie. C'est un débat difficile, chacun connaît les positions de nos partenaires, mais je pense que personne ici ne peut accepter que les prix de production de l'électricité en France, qui sont modérés grâce aux choix énergétiques que nous avons faits depuis les années 1960, soient directement affectés par l'augmentation des prix du gaz, et que le coût marginal d'augmentation d'une centrale à gaz dans l'est de l'Europe définisse le prix de l'électricité produite dans une centrale nucléaire en France.

réservée à chaque personne ayant un revenu inférieur à 2 000 euros. De ce point de vue, je tiens à dire que nous regrettons, avec Olivier Dussopt, que vous ayez supprimé cette mesure simple et rapide qui concerne 38 millions de personnes et qui permet d'apporter une protection contre l'augmentation des prix pour toute personne, je le répète, ayant un revenu inférieur à 2 000 euros. Votre mesure de remplacement, que j'ai évidemment étudiée soigneusement, exclut les retraités et les indépendants. Non ! Je considère donc qu'elle est moins juste et moins efficace. Par conséquent, la majorité rétablira en nouvelle lecture notre proposition initiale d'indemnité inflation pour chacun de nos compatriotes qui a un revenu inférieur à 2 000 euros. C'est la protection que nous devons à nos compatriotes face à l'augmentation des prix.

Je vois trois sujets majeurs sur lesquels le projet de loi de finances s'engage et qui doivent nous permettre de poursuivre sur la voie du redressement économique de notre pays et de renouer avec des performances économiques du meilleur niveau et- enfin ! -avec un plein-emploi que nous n'avons pas connu depuis un demi-siècle. Le premier Le premier défi, c'est la réduction du chômage et des inégalités. Ce combat, nous commençons à le gagner, mais la partie qui reste devant nous est la plus difficile, parce que, pour arriver enfin au plein-emploi que beaucoup de nos partenaires européens et occidentaux connaissent, pour sortir d'un demi-siècle de chômage de masse qui a fragilisé la société française tout entière, il faut poursuivre dans la voie d'un certain nombre de politiques qui sont courageuses et difficiles, mais qui donnent des résultats. Réformer l'assurance chômage, lorsqu'il y a des propositions d'emplois qui se multiplient, qu'on a créé un million d'emplois en cinq ans, 500 000 au cours des dernières années, est une question d'efficacité et de justice. Il est légitime de réformer l'assurance chômage, d'augmenter le nombre de mois de cotisations avant d'avoir accès à une indemnisation et d'être très strict sur le respect des règles. Il existe des règles pour pouvoir bénéficier d'une indemnisation du chômage.

Il faut également, en début de carrière professionnelle, multiplier les dispositifs qui permettent de développer l'apprentissage. Nous sommes en train de gagner cette bataille de l'apprentissage que beaucoup d'entre vous souhaitaient voir livrée depuis des années. Nous sommes en train de devenir une grande nation d'apprentis. L'apprentissage, on le sait tous, c'est la meilleure voie d'entrée sur le marché du travail. C'est celle qui a été employée par nos partenaires allemands avec efficacité, et c'est celle que nous avons développée. Il faut poursuivre dans cette voie, car elle donne des résultats, d'autant que toutes les entreprises, même les plus petites, jouent parfaitement le jeu.

Le véhicule thermique se transformant progressivement en véhicule électrique, l'industrie automobile connaît la révolution technologique et industrielle la plus importante depuis le début du XX siècle. Aussi, il va falloir accompagner des dizaines de milliers de salariés pour leur permettre d'acquérir une nouvelle formation, une nouvelle qualification. On doit pouvoir dire à chaque ouvrier qui travaille aujourd'hui dans une fonderie, et qui sait parfaitement que le volume de commandes va diminuer- il y a quatre fois moins de pièces de fonte dans un moteur électrique que dans un moteur diesel ou essence -, que l'on va lui donner une nouvelle formation et l'accompagner vers un nouvel emploi.

Enfin, pour gagner définitivement cette bataille du chômage, il faut évidemment engager une réforme des retraites, de sorte que nous ayons un âge légal de départ à la retraite plus tardif pour tenir compte de l'allongement de la durée de la vie, chacun étant incité à travailler plus longtemps.

Cela suppose des investissements supplémentaires dans le nucléaire, avec l'ouverture de nouveaux réacteurs, comme l'a annoncé le Président de la République, l'investissement dans des réacteurs de nouvelle génération, le financement d'installations pour l'hydrogène vert, toutes choses que nous avons déjà engagées. Je veux souligner à quel point ce défi est difficile à relever et demande beaucoup de constance dans nos choix. Surtout de la constance d'Ascoval, une entreprise que nous avons sauvée dans le nord de la France. Cette aciérie est confrontée aujourd'hui, alors qu'elle est parfaitement rentable, à une augmentation du prix des matières premières et de l'électricité. Nous avons apporté une première réponse à cette entreprise au travers d'un amendement voté à l'Assemblée nationale pour toutes les entreprises fortement consommatrices d'énergie. Celui-ci prévoit une compensation financière

Nous avons ensuite fait le choix d'engager des dépenses massives pour protéger les salariés et des entreprises. L'Institut des politiques publiques vient de l'indiquer très clairement, il était moins coûteux de dépenser de l'argent pour protéger les salariés, éviter l'explosion du chômage et les faillites de masse, que de laisser faire et d'avoir une crise économique et sociale avec, derrière, des coûts absolument considérables. Nous avons une dette de 115 % au moment où je vous parle ; elle aurait été, selon cet institut, de 126 % si nous n'avions pas dépensé d'argent public pour protéger les salariés et les entreprises. Nous continuerons à le faire, car la réduction de la dette, progressive et déterminée, est un impératif pour la Nation. Cela passe par de la croissance ; cela passe également par les réformes que j'ai indiquées- assurance chômage et réforme des retraites cela passe enfin par un budget adopté sous une forme pluriannuelle, de façon à avoir de la visibilité et un calendrier clair sur la réduction de cette dette. La parole

Madame la présidente, monsieur le ministre- cher Bruno Le Maire -, monsieur le président de la commission des finances, monsieur le rapporteur général, mesdames, messieurs les sénateurs, dans le contexte macroéconomique brossé par le ministre de l'économie à l'instant, nous avons préparé un projet de loi de finances pour 2022

C'est la raison pour laquelle le budget que nous vous présentons prévoit de revaloriser un certain nombre de budgets, en commençant par les crédits accordés aux fonctions régaliennes de l'État.

De la même manière, nous vous proposons d'augmenter le budget du ministère de la justice de 8 % pour la deuxième année consécutive, soit une augmentation de crédits de 670 millions d'euros. Ainsi, en 2022, nous aurons non seulement rattrapé la trajectoire de la loi de programmation pour la justice, mais nous serons même au-delà, avec une exécution à laquelle nous veillons, et qui a été l'objet de discussions, hier, à l'occasion de l'examen du projet de loi de finances rectificative.

dont 200 millions d'euros seront consacrés au financement par l'État de la participation obligatoire des employeurs publics à la protection sociale complémentaire, à l'instar de ce que nous avons prévu pour tous les ministères.

et pour financer les mesures en faveur de la vie étudiante. Je pense notamment à la revalorisation des crédits consacrés aux bourses du fait de l'augmentation du nombre d'étudiants boursiers, mais aussi à des mesures d'accompagnement de la sortie de crise. Préparer l'avenir, c'est aussi anticiper et accompagner la transition écologique. À cette fin, le budget du ministère de la transition écologique augmentera de 1,5 milliard d'euros,

nous vous proposons de mettre en oeuvre un engagement pris devant vous par ma collègue Sophie Cluzel, consistant à prévoir un abattement sur les revenus des bénéficiaires de l'AAH vivant en couple. Cela permettra à 110 000 allocataires de bénéficier d'une revalorisation de 110 euros par mois. domaine de la solidarité, nous voulons maintenir notre effort en matière de lutte contre les discriminations et en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes. Le total des crédits consacrés à cette thématique, lorsque l'on agrège tous les ministères, s'élève à 1 milliard d'euros. Les crédits pilotés directement par le ministère délégué à l'égalité entre les femmes et les hommes sont plus modestes- ils financent le 39 19, qui est désormais ouvert sept jours sur sept, et différents appels à projets. Ils s'élevaient à 28 millions d'euros voilà deux ans et seront de 51 millions d'euros cette année. Par

la dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) est reconduite à hauteur de 1 milliard d'euros ; la dotation de soutien à l'investissement local (DSIL) est, elle aussi, reconduite à hauteur de 1 milliard d'euros, que nous allons revaloriser de 350 millions d'euros supplémentaires, avec la volonté de flécher principalement cette somme sur les projets inscrits dans les contrats de relance et de transition écologique, dont nous souhaitons la signature avec les intercommunalités.

Nous vous proposons donc la stabilité, avec la mise en oeuvre d'une tranche supplémentaire de suppression de la taxe d'habitation, ce qui ne change pas désormais le panier de ressources des collectivités. C'est aussi au nom de cette stabilité

sont les priorités que nous finançons, et nous le faisons en respectant trois lignes directrices en matière budgétaires. La première ligne directrice ne vous surprendra pas, puisque c'est celui que nous suivons depuis le début du quinquennat

de ne pas inscrire dans ce projet de loi de finances des mesures extrêmement structurées et dures, qui auraient peut-être été de nature à accélérer le redressement des finances publiques, nous continuons à moderniser et à simplifier à chaque fois que nous le pouvons. Notre volonté est d'accompagner la relance de la croissance, car c'est ce qui va nous permettre de faire face à nos engagements financiers. Nous ne voulons pas répéter l'erreur de vouloir redresser trop rapidement les comptes publics, au risque d'étouffer la croissance. C'est la raison pour laquelle nous sommes plutôt sur une voie de normalisation.

Hors dépenses consacrées au plan de relance et hors reste à payer consacré aux mesures d'urgence, les dépenses dites ordinaires de l'État sont donc maintenues et maîtrisées. nous vous proposons un projet de loi de finances qui s'appuie sur une hypothèse d'évolution des dépenses publiques hors relance et hors urgence, toutes administrations confondues, à 1 % en volume, ce qui est aussi le signe et l'illustration d'une forme de normalisation en matière de finances publiques. quels sont les résultats que nous vous proposons d'atteindre avec ce projet de loi de finances ? Nous voulons d'abord respecter l'engagement que nous avons pris devant vous de décrue progressive du déficit public. Nous étions à 9,1 % en 2020,

à diminuer le déficit. Dans ces conditions, peut-être pourrions-nous espérer atteindre 8 %, voire 7,9 %. Enfin, nous serons sur un déficit égal ou inférieur à 5 % en 2022, ce qui est la marque d'une trajectoire de redressement et l'annonce d'un retour à une situation, qui, si elle reste dégradée, nous paraît un peu plus normale et soutenable. Le niveau de la dette sera lui aussi moins important que prévu, comme je l'ai indiqué hier. Nous prévoyons pour 2022 une dette représentant 113,5 % du PIB, alors qu'il y a quelques mois encore nous craignions d'atteindre les 120 %. Le poids de la dépense publique par rapport au PIB sera également revu à la baisse, à hauteur de 56 % à 57 %, ce qui correspond peu ou prou au niveau de 2018. Je rappelle que nous avions atteint 53,5 % en 2019. C'était également l'un des engagements qui avaient été pris.

Madame la présidente, messieurs les ministres, monsieur le président de la commission des finances, mes chers collègues, l'an dernier, à la même place, nous ouvrions l'examen du projet de loi de finances dans le contexte d'un reconfinement de la France et du retour à grande force du virus de la covid-19. Cette année, alors que la reprise économique s'avère plus forte que nous l'avions espérée au cours des derniers mois, c'est un budget livré « en kit » que nous nous apprêtons à discuter. discuter. Lors de son dépôt, le 22 septembre, il a même été qualifié d'incomplet par le Haut Conseil des finances publiques lui-même, dans la mesure où les principales mesures annoncées au cours des derniers mois, à savoir, notamment, le grand plan d'investissement, devenu France 2030, et le revenu d'engagement, devenu contrat d'engagement jeune, n'y figuraient pas. Depuis, au gré des déplacements présidentiels et ministériels, de nouvelles annonces se font jour, se concrétisant, pour la plupart d'entre elles, dans le projet de loi de finances au fil de son examen à l'Assemblée nationale. D'un budget incomplet, nous sommes passés, autant le dire, à un budget de campagne, assorti de mesures pour le moins hétéroclites. Il y en a pour tout le monde, ou presque ! Pour cela, l'exécutif profite d'une embellie économique inespérée, puisque la croissance pour 2021 pourrait atteindre plus de 6,6 %, et même 6,8 %- monsieur le ministre, je suis plutôt d'accord avec vous sur ce point. L'ampleur de la reprise en 2021 constitue évidemment une bonne nouvelle et elle offre une rampe de lancement particulièrement favorable pour l'économie en 2022. Ainsi, dans l'hypothèse pessimiste où l'activité ne progresserait pas au cours du quatrième trimestre, l'acquis de croissance en 2022 pourrait s'élever à 1,8 %, niveau qui n'a été dépassé que trois fois en trente Pour autant, les conjoncturistes jugent que la prévision de croissance à 4 % en 2022 est optimiste, sachant que la forte croissance en 2021 témoigne davantage d'un rattrapage plus précoce que d'une amélioration de nos fondamentaux économiques.

auparavant crédibles, sont désormais dépassées, au moins pour 2021, avec une inflation de l'indice des prix à la consommation harmonisé de 2 %, contre 1,7 % prévu. % prévu. L'éventuelle poursuite de la hausse des prix de l'énergie pourrait réduire la croissance en pesant non seulement sur la consommation des ménages, mais aussi sur la compétitivité des entreprises.

Il faut, par ailleurs, garder à l'esprit que la question des prix de l'énergie s'articule avec l'augmentation tendancielle des prix des matières premières et des difficultés de recrutement : autant de facteurs qui ont un impact sur les prix de vente et donc sur l'inflation ou sur la profitabilité et la compétitivité des entreprises. Enfin, une reprise importante de l'épidémie de covid-19 ne serait, bien sûr, pas sans conséquence. Face à ces aléas, le Gouvernement a apporté une réponse au fil de l'eau, en direction des ménages et des fournisseurs d'électricité. S'agissant de l'état de nos finances publiques, je ne cache plus mon inquiétude. Depuis le début de l'épidémie, nous avons été soucieux de donner au Gouvernement les moyens d'agir dans l'urgence face à la crise, ainsi que pour la relance. Un volume important de dépenses ou de baisses de recettes a été autorisé pour soutenir notre économie, ce qui n'a pas été un mauvais choix : au sortir de la crise, nos capacités de production ont été préservées. situation extraordinaire ne saurait avoir ni effacé la mémoire de notre commission ni exonéré le Gouvernement de toute responsabilité en matière de maîtrise des comptes publics. Ainsi, contrairement à ses engagements pris en loi de programmation et à l'effort assez ambitieux qu'il s'était assigné, le Gouvernement a abandonné tout effort de maîtrise des dépenses à compter de 2019. Concrètement, ce relâchement signifie que les dépenses primaires ont poursuivi une trajectoire de hausse très importante tout au long du quinquennat, avec une croissance en volume de l'ordre de 1,2

Compte tenu du scénario de croissance et des dépenses nouvelles qui s'ajoutent à ce qui était prévu initialement dans le projet de loi de finances, le solde public atteindrait donc 5 % du PIB en 2022, avec un taux d'endettement de 113,5 %. particulièrement critiquable le fait que 40 milliards d'euros de dépenses primaires soient à ce jour constatés. La dernière fois que nous avions pu assister à une hausse de cette ampleur, c'était en 2017, à l'aube- est-ce une surprise ? -d'une autre campagne présidentielle. Quoi qu'il en soit, le Gouvernement n'a pas voulu mettre à profit les bénéfices d'un regain inattendu de la croissance pour réduire notre endettement et assainir nos finances publiques. J'observe que, parallèlement, les administrations publiques locales produisent, elles, les efforts demandés. Leurs dépenses de fonctionnement augmenteraient ainsi seulement de 0,9 % en volume en 2022, ce qui signifie qu'elles auraient progressé de 1,1 % en moyenne depuis 2019. Avouez, messieurs les ministres, que c'est un effort substantiel et méritoire de maîtrise des dépenses de la part des collectivités territoriales, dans la mesure où, sur une longue période, ces dépenses croissent tendanciellement d'environ 1,9 % par an en volume. La stratégie affichée du Gouvernement en matière de maîtrise des comptes publics pour l'avenir ne laisse pas de m'inquiéter. Il propose en effet de limiter la croissance annuelle de la dépense primaire hors mesures d'urgence et de relance à 0,4 % par an en volume entre 2022 et 2027. Un tel résultat serait empiriquement inédit, et je ne peux que redire combien il nécessite, pour être crédible, de déterminer et de présenter les moyens envisagés pour y parvenir. Or une telle documentation

D'ailleurs, en pratique, le Gouvernement s'était déjà engagé sur un objectif comparable en début de quinquennat. Il réitère donc aujourd'hui une promesse qu'il n'a pas su tenir. su tenir. Devant l'absence de résultats, la trajectoire proposée par le Gouvernement s'apparente, de mon point de vue, à une simple mesure d'affichage. La crise sanitaire ne peut masquer ni le manque de sérieux budgétaire du Gouvernement au cours du quinquennat ni l'absence de perspectives crédibles d'amélioration des comptes publics. la maîtrise de la dépense publique et l'assainissement de nos comptes publics sont une nécessité absolue. Il y a une véritable urgence à transformer la simple promesse en un véritable engagement. S'agissant plus précisément du budget de l'État, après un niveau inédit en 2021, avec un déficit de 205 milliards d'euros, selon les prévisions du projet projet de loi de finances rectificative de fin d'année, le budget 2022 affiche désormais un déficit qui reste particulièrement élevé, à 155,1 milliards d'euros, dont près de 12 milliards supplémentaires sous le seul effet des mesures adoptées par l'Assemblée nationale, tant en recettes, avec le bouclier tarifaire, qu'en dépenses. Le Gouvernement semble donc considérer que le niveau de déficit atteint au plus fort de la crise de 2009 et 2010 est désormais, en quelque sorte, un régime de croisière normal pour le paquebot de l'État. Or ce paquebot s'alourdit d'une dette qui ne cesse de croître et de s'aggraver, avec des émissions nouvelles de 260 milliards d'euros pour la troisième année consécutive.

tout le niveau. Le déficit n'est pas dû aux recettes, qui bénéficient, elles, de la reprise économique. Le bouclier tarifaire introduit par amendement à l'Assemblée nationale réduit toutefois ces recettes de 5,3 milliards d'euros, mais cela sera certainement davantage, puisque ce chiffre a déjà été révisé à 5,9 milliards d'euros. Le projet de loi de finances n'introduit pas de réforme fiscale de grande ampleur et se place dans la continuité des années précédentes. Sur l'ensemble du quinquennat, le niveau global des recettes fiscales nettes est stable, autour de 290 milliards d'euros, et on peut observer un choix marquant du Gouvernement à transférer de plus en plus de parts de fiscalité à des tiers, tels que la sécurité sociale ou les collectivités : ainsi, la fiscalité affectée est désormais de 335 milliards d'euros et dépasse le le montant des recettes fiscales revenant à l'État lui-même. Par conséquent, le surcroît des recettes qui résulterait de la croissance ne profiterait que partiellement à l'État, ce qui rendra le remboursement de la dette encore plus difficile. C'est donc aux dépenses que le déficit est dû à titre principal. Le sujet est pour le moins mouvant, compte tenu des 277 amendements que l'Assemblée nationale a adoptés en seconde partie de la loi de finances, dont 113 présentés par le Gouvernement. Autant le budget déposé en septembre était famélique et incomplet, autant celui qui nous est transmis porte des mesures de dépenses en surabondance. Rendez-vous compte : hors missions « Plan de relance » et « Plan d'urgence », les dépenses dites pilotables étaient, dès le dépôt du texte en septembre, donc avant les mesures nouvelles, en augmentation de 11,8 milliards d'euros, soit 4,1 %, à périmètre constant, par rapport à la loi de finances initiale pour 2021. Les dépenses courantes continuent la progression qui a marqué l'ensemble du quinquennat, loin, très loin des objectifs de diminution fixés voilà quatre ans. Nous assistons là à une véritable dérive. Et la quasi-totalité des missions du budget général est concernée par les augmentations de dépenses. Il y en a vraiment pour tout le monde ! Le plus marquant est bien sûr l'amendement, inédit sous la V République par son montant, qui ouvre 34 milliards d'euros d'autorisations d'engagement pour le plan d'investissement France 2030, dont nous ignorons toutes les modalités, et qui pèse déjà à hauteur de 3,5 milliards d'euros sur le solde en 2022. Cet amendement est l'exemple même des mesures qui, prises en toute fin du quinquennat, augmentent les engagements de l'État et instaurent une contrainte à la hausse sur les dépenses des prochaines années et pour le prochain président de la République. S'agissant enfin des emplois, 850 équivalents temps plein sont créés dans les ministères au titre des missions du budget général. Toutefois, le Gouvernement a réduit artificiellement les plafonds d'emplois de près de 7 000 équivalents temps plein travaillés en excluant tout simplement les apprentis de leur décompte. Sur l'ensemble du quinquennat, le nombre d'emplois est stable, le Gouvernement ayant totalement abandonné l'objectif initialement fixé d'une baisse de 50 000 emplois, tandis que la masse salariale poursuit inexorablement son augmentation. En conclusion, la commission des finances a proposé d'adopter la première partie de ce projet de loi de finances, sans entrain et avec un nombre limité d'amendements techniques et de correction des dispositifs qui lui étaient transmis par l'Assemblée nationale. Je lui proposerai demain matin, en complément, d'adopter deux amendements, déjà annoncés, qui me paraissent devoir être présentés du fait de l'importance de leurs sujets. Le premier concerne les collectivités locales, car j'estime nécessaire de prévoir une compensation intégrale des entreprises (CVAE), estimée à 5 % en 2022. Il s'agit là non seulement d'une conséquence de la crise, du fait de la mécanique de cette cotisation, mais aussi d'une forme de reconnaissance et d'un juste retour de l'action et de la présence des collectivités territoriales, en première ligne pendant la crise. Le second vise à s'attaquer à la fraude, puisque je proposerai un renforcement du dispositif de lutte contre les arbitrages de dividendes, pratique mise en lumière par l'affaire des « » en 2018 et contre laquelle la commission des finances avait déjà présenté un amendement.

Cela nous a conduits à proposer de ne pas adopter les crédits de plusieurs missions et comptes d'affectation spéciale. Ainsi peuvent être résumés les résultats des travaux de la commission des finances avant d'aborder l'examen en séance d'un budget à la fois évolutif et manifestement tourné vers la prochaine campagne présidentielle, dont il porte très clairement la marque. La parole

Comme il est de tradition, je rappellerai qu'il succède à plusieurs semaines d'analyse approfondie du volet budgétaire et fiscal de ce texte en commission, depuis sa présentation en Conseil des ministres le 22 septembre dernier. Le rapporteur général, les rapporteurs spéciaux et les rapporteurs pour avis ont conduit un nombre considérable d'auditions pour se forger une opinion sur tous les aspects de ce budget, et je veux saluer leur engagement à l'ouverture de nos débats. Cet engagement est d'autant plus méritoire que, dès l'origine, il nous a été indiqué que le budget 2022 serait complété « au fur et à mesure » des arbitrages présidentiels sans considération du temps nécessaire aux parlementaires pour évaluer les mesures nouvelles soumises à leur vote. L'Assemblée nationale a ainsi été invitée à ouvrir pas moins de 34 milliards d'euros de crédits pour le plan France 2030 par voie d'amendement, un mois et demi après la présentation du projet de loi de finances, sans étude d'impact et avec une idée très schématique de la manière dont ils seront dépensés. Faites-nous confiance »- cela me rappelle la chanson du, « Confiance, aie confiance ... »-semble nous dire le Gouvernement, considérant manifestement qu'il n'appartient pas aux parlementaires d'examiner sérieusement l'opportunité d'engager ces dépenses.

Au-delà de ce rappel de principe, j'en viens aux caractéristiques essentielles de ce projet de loi de finances, telles qu'elles apparaissent aujourd'hui. Tout d'abord, ce budget est marqué par le retour bienvenu de la croissance, avec une estimation à hauteur de 4 % en 2022, après une croissance qui pourrait atteindre 6,75 % à 6,8 % cette année, si l'on en croit les dernières prévisions de la Banque de France. Certes, le PIB a fortement chuté en 2020 et retrouve tout juste son niveau de 2019, mais chacun pourra se réjouir du redémarrage de l'économie, même si celui-ci reste soumis à de nombreux aléas tant sanitaires qu'économiques

en ne mettant pas fin brutalement au soutien budgétaire, qui a d'ailleurs en partie contribué à l'alimenter, et, d'autre part, à ne pas laisser de côté certains de nos concitoyens. La hausse des prix de l'énergie et plus généralement le retour de l'inflation pèsent sur le budget des ménages les plus modestes, ce qui justifie un accompagnement ciblé, qui doit aller au-delà d'une aide ponctuelle. À cet égard, l'indemnité inflation relève plus d'une solution ponctuelle que d'une réponse construite au défi posé par une hausse des prix qui risque de se poursuivre en 2022.

La crise que nous avons traversée a aussi eu des répercussions très fortes sur la jeunesse. Le contrat d'engagement jeune qui se substituerait à la garantie jeunes pour environ 400 000 jeunes sans emploi ni formation ou études n'est pas à la hauteur des enjeux, comme nous le savons tous.

Le budget 2022 voit la plupart des missions budgétaires augmenter, ce qui ne surprend guère en période préélectorale. Le déficit s'établirait encore à 5 % du PIB en 2022, bien au-dessus de l'objectif de 3 %, et la dette s'élèverait à 113,5 % du PIB.

après l'élection présidentielle, « d'entreprendre un rééquilibrage progressif mais global des finances publiques » pour réduire son endettement. Et le FMI de considérer que « la poursuite des réformes déjà prévues, telles que celles des retraites, de l'assurance chômage et de la fonction publique, contribuerait considérablement au rééquilibrage nécessaire ». Je regrette que ces préconisations sur les seules dépenses, qui rejoignent d'ailleurs celles de la Cour des comptes, omettent le fait qu'un budget résulte toujours d'un équilibre entre recettes et dépenses. Le ministère des finances a lui-même calculé que ce quinquennat se sera traduit par près de 50 milliards d'euros d'allègement de la pression fiscale, dont la moitié sur les ménages et l'autre sur les entreprises.

des impôts de production, dont nous ne partageons pas la philosophie. Récemment, France Stratégie, confirmant les analyses que nous avions faites,

Nous sommes loin du « ruissellement » promis- si les services du Premier ministre le disent eux-mêmes, comment ne pas les croire ? Enfin, malgré les annonces de l'OCDE, tout reste encore à construire en matière d'imposition des multinationales,

d'une part, de mettre fin au « désarmement fiscal » auquel il a été procédé au cours de ce quinquennat, afin de renforcer l'équité entre les citoyens et entre les générations ; d'autre part, de préparer l'avenir en veillant à ne pas sacrifier les dépenses durablement favorables à la croissance économique, au progrès social et environnemental, dans la lignée de la position exprimée par la Commission sur l'avenir des finances publiques. Nous passons

Madame la présidente, messieurs les ministres, mes chers collègues, nous voici arrivés au jour de l'ouverture de l'examen du projet de loi de finances pour 2022. Il s'agira du dernier budget du quinquennat de M. Macron, aussi nous paraît-il judicieux de tirer un bilan global de ces cinq années. Nos collègues de la majorité sénatoriale eurent, il y a quelques semaines de cela, des mots très durs à l'endroit du présent budget. Voici, en effet, ce que vous déclariez, mes chers collègues : « Le Gouvernement n'envisage plus le projet de loi de finances que comme un bout de torchon et il ajoute ensuite des mesures au fur et à mesure. Mais la réponse est non. Ce n'est pas comme cela qu'on gère la France. » J'ajoute cette seconde déclaration C'est vrai qu'on peut se poser la question de savoir si cela vaut la peine de perdre trois semaines pour corriger les imperfections d'un budget indécent ». Notre groupe, lors de la discussion générale, déclinera ses propositions par la voix de nos collègues, Pascal Savoldelli, d'une part,

C'est une étude récente de France Stratégie qui nous le dit. Le ruissellement annoncé ne s'est pas produit. Par contre, les revenus des 0,1 % les plus riches de notre pays ont explosé. Or cette mesure était censée « favoriser la croissance de notre tissu d'entreprises, stimuler l'investissement et l'innovation ».

Si la fortune des 500 premiers milliardaires a crû de 30 %, celle des cinq premiers a grimpé de 45 % ! L'instauration du prélèvement forfaitaire unique a incontestablement eu des effets, puisqu'elle a entraîné une hausse de 60 % des dividendes distribués,

De plus, l'étude précitée indique que cette augmentation des dividendes est de plus en plus concentrée sur la population. En 2018, 0,1 % des foyers fiscaux, soit 38 000 personnes environ, ont perçu les deux tiers des montants totaux et les ultrariches, soit 0,01 % des foyers fiscaux ou 3 800 qui en captaient un cinquième, en ont reçu le tiers. Tel est, mes chers collègues, le bilan vu du côté des patriciens ; tournons-nous désormais du côté des plébéiens. Voyons où en est la France des fins de mois difficiles, celle où la moindre dépense imprévue peut faire basculer dans la précarité. Dans notre pays, en effet, un Français sur cinq a du mal à joindre les deux bouts. Est considéré comme pauvre celui dont le niveau de vie est inférieur au seuil de pauvreté, fixé à 60 % du niveau de vie médian, soit aujourd'hui 1 063 euros pour une personne seule, à un peu moins de 200 euros du montant net du SMIC quand on y songe, mes chers collègues ... Pas moins de 14,6 % de la population survit dans ces conditions. Au-delà des statistiques froides, ce sont des situations humaines difficiles, parfois dramatiques, qu'il nous faut considérer. Un tiers de la population française puise dans ses économies pour boucler son budget et la moitié se déclare au moins en difficulté de logement, selon l'Insee. En France, 2,3 millions de personnes vivent avec au mieux 735 euros par mois pour une personne seule 4 millions de ménages doivent se contenter de minima sociaux, ce qui représente plus de 6 millions de personnes si l'on inclut les conjoints et les enfants. Il y a aussi toutes celles et tous ceux qui connaissent l'insécurité alimentaire. Cette année, 5 millions de nos concitoyennes et concitoyens ont eu recours à l'aide alimentaire. La Fondation Abbé Pierre indiquait, dans un rapport publié la semaine dernière, que deux Français sur dix ont froid chez eux. Certains allument le chauffage quand la température des chambres tombe sous les 14 degrés. Les 20 % des ménages les plus modestes consacrent 16 % de leurs revenus aux dépenses énergétiques, quand pour les 20 % des ménages les plus aisés le chiffre tombe à 4,5 %. Certes, le Gouvernement se targue d'avoir rendu 24 milliards d'euros aux ménages. Il nous faut analyser ces données avec beaucoup de précision. En valeur absolue, ce sont bien les ménages les plus aisés qui ont bénéficié de ces gains,

Précarité et pauvreté restent à un niveau très élevé dans notre pays. Peu de personnes arrivent à en sortir durablement et une partie importante de la population éprouve de plus en plus de difficultés à faire face aux dépenses courantes. Au surplus, la plupart du temps, les améliorations proviennent d'opérations reposant sur des primes ou des exonérations quand la vraie réponse passerait par une hausse durable et sensible des salaires et des pensions. Comment s'étonner, dans ce contexte, que la question des salaires et du pouvoir d'achat soit devenue la première préoccupation de nos concitoyens ? Or vous choisissez ce moment pour mettre en oeuvre la réforme de l'assurance chômage, en vue de réaliser des économies budgétaires ! Votre saupoudrage de mesures ne peut suffire à constituer une réponse efficace à la problématique du pouvoir d'achat. L'augmentation des prix de l'énergie et le léger sursaut d'inflation inquiètent légitimement le pays. Ainsi, 56 % des Français estiment que leur pouvoir d'achat a plutôt diminué sous la présidence de M. Macron. Entre des classes moyennes et populaires insatisfaites, à 64 % et 56 % respectivement, et des classes aisées qui le sont bien moins, à seulement 19 %, l'image du « président des riches » est un véritable sparadrap. À l'évidence, il n'y a pas eu dans ce quinquennat de réelle volonté de s'attaquer aux profondes inégalités qui traversent notre société. Les laisser ainsi s'accroître, c'est courir un très grand risque social et politique. Oui, nous restons convaincus que l'impôt juste, équitable et progressif est une arme efficace contre ces problèmes. Nous pensons utile de rétablir un ISF rénové et renforcé. À celles et ceux qui disent que ce n'est pas avec cette seule mesure que l'on va redresser la France, nous rappellerons que les 5,2 milliards d'euros de recettes que cet impôt produisait avant sa suppression sont à mettre en regard des budgets présentés dans ce projet

Cela a commencé avec la réforme de l'assurance chômage. Emmanuel Macron, président-candidat ou candidat-président, a déjà donné des gages aux libéraux sur « l'incontournable » réforme des retraites, qu'il mettrait en oeuvre, dit-il, dès 2022 ... Nous voilà tous prévenus ! Pour ce dernier budget du quinquennat, les choix attendus par le pays n'ont à l'évidence pas été faits. Vous n'abandonnez pas le dogme de la baisse draconienne des dépenses publiques, prévue dans le cadre du programme de stabilité, puisque celle-ci constitue la contrepartie aux réductions d'impôts qui profitent aux plus fortunés de nos concitoyens.

pour que les Seychelles soient retirées de la liste des paradis fiscaux ... Toujours cette ambivalence qui illustre le manque d'une véritable volonté politique du Gouvernement de s'attaquer radicalement à ce scandale de notre temps ! Pourtant, les sommes en cause dans ces différentes révélations sont absolument vertigineuses. Votre action, globalement, s'apparente davantage à un saupoudrage cosmétique qu'à une intervention en profondeur. Ce budget devrait mobiliser les crédits nécessaires aux grands investissements de la transition écologique. La récente COP26 de Glasgow a montré à quel point des moyens financiers considérables devaient être engagés. Consacrer 10 milliards d'euros par an à la rénovation des bâtiments publics et des logements permettrait par exemple de réduire la consommation énergétique des ménages, donc leur facture. Cinq années après le vote du premier budget de votre quinquennat,

question préalable est une idée qui a traversé l'esprit de plusieurs de nos collègues de la majorité sénatoriale. Il ne s'agit pas de faire l'école buissonnière ; notre groupe soumet donc cette motion au débat. C'est toute la logique de cette construction budgétaire qu'il convient de rejeter.

amélioré la vie de millions d'entre eux qui cherchaient un travail, qui en ont trouvé et qui bénéficient, à l'heure où je vous parle, d'une meilleure rémunération que celle dont ils pouvaient disposer au début du quinquennat.

nous voulons le faire par l'éducation, la formation et la qualification. Vous croyez à une redistribution toujours plus forte dans un pays dont le taux d'imposition est le plus élevé

où le taux de prélèvements obligatoires est le plus élevé de tous les pays développés. Si les impôts faisaient le bonheur des gens, nous serions la Nation la plus heureuse de la planète ; ce n'est pas le cas. cas. Je conteste donc votre proposition politique, car j'estime que c'est la voie qui a été empruntée pendant des décennies et des décennies, et qui a contribué au malheur français. Quand vous retirez à ceux qui travaillent une trop grande partie du produit de ce travail, ne vous étonnez pas que le désespoir,

et les drames sociaux partout en France. Aucune autre majorité n'a eu le courage d'investir autant d'argent dans l'activité partielle pour éviter un drame social ou politique et pour faire en sorte de protéger l'emploi dans notre pays ! Telle est notre ligne conductrice : le travail, le travail, le travail. Et du travail qui paie-

la défiscalisation des heures supplémentaires, la défiscalisation des pourboires, la suppression de la taxe à 20 % sur l'intéressement et sur la participation, tout cela permet de mieux associer les salariés aux résultats de l'entreprise, de sorte qu'un salarié rémunéré au niveau du SMIC pourra toucher non pas 1 270 euros net par mois, mais presque 1 500 euros. Certains candidats de la droite en ont rêvé, nous l'avons fait pendant ce quinquennat, près de 1 500 euros net par mois grâce aux aides de l'État, car nous croyons au travail qui paie. Il est vrai, effectivement, qu'à nos yeux il est bon que les Français gardent une partie du produit de leur travail et que tout ne leur soit pas pris par les impôts.

nous ne voterons pas la question préalable.

demande plus à voter ? ... Le scrutin est clos.

est pour nous une étape incontournable de la vie parlementaire et, à travers elle, de la vie démocratique du pays. Ce projet de loi de finances pour 2022 n'échappe évidemment pas à cette règle.

L'intervention massive de l'État, en 2020 et 2021, pour soutenir le tissu productif et le tissu social, pour préserver nos entreprises d'une vague de faillites et leurs salariés du chômage,

Mais ce soutien de l'État, nécessaire durant la crise- nous l'avons d'ailleurs soutenu plusieurs projets de loi de finances rectificative -, s'est immanquablement traduit par une dégradation importante des ratios de finances publiques. S'il est inévitable que la dette publique augmente dans de telles proportions en période de crise et de récession, il nous paraît désormais indispensable d'en reprendre le contrôle pour en assurer la soutenabilité. Nous devons donc nous fixer un cap pour accélérer la décrue du déficit public, de façon à stabiliser dès que possible le poids de la dette par rapport à notre produit intérieur brut. nous sommes convaincus qu'une croissance vertueuse y pourvoira. Une lutte plus efficace contre la fraude et l'évasion fiscales pourrait aussi y contribuer. Notre groupe fera des propositions en ce sens ; nos collègues Sylvie Vermeillet et Michel Canévet auront l'occasion d'y revenir dans un instant. Très bien ! De même, la bonne tenue de l'investissement privé ne doit pas faire oublier l'impératif de justice fiscale. C'est pourquoi le groupe Union Centriste vous proposera de supprimer une niche fiscale implicite sur la transmission du nouveau plan d'épargne retraite issu de la loi Pacte,

à 30 %, même si plusieurs facteurs expliquent ce résultat. La première partie de ce projet de loi de finances, dont nous entamons aujourd'hui l'examen, ne contient au bout du compte qu'une seule mesure fiscale nouvelle d'un montant significatif, le bouclier tarifaire en matière d'énergie. Le gel des tarifs réglementés du gaz, le plafonnement de l'augmentation des tarifs réglementés de l'électricité, le rehaussement du chèque énergie pour 6 millions de ménages et le complément prévu dans le dernier PLFR forment un bloc indispensable pour préserver autant faire se peut le pouvoir d'achat des Français dont les revenus sont les plus modestes. concerne plus particulièrement les collectivités locales, qui contribuent activement, on le sait, à la vie des territoires, il est indispensable de maintenir leur capacité à investir.

: hausse de la péréquation de 190 millions d'euros en faveur des communes, doublement des crédits affectés à la dotation de soutien aux communes pour la protection de la biodiversité et la valorisation des aménités rurales, désormais ouverte aux communes membres d'un parc naturel régional,

La réduction du taux d'imposition sur les bénéfices des sociétés, destinée à renforcer l'attractivité de notre pays, s'est aussi poursuivie, malgré quelques contretemps budgétaires en début de législature puis au moment du mouvement des gilets jaunes.

enfin, dans le cadre du plan de relance lancé à la fin de l'année dernière, la baisse des impôts dits de production, qui figurait également dans les cartons de l'exécutif. Cette dernière mesure n'est pas sans conséquence sur les finances des collectivités locales

qui nécessite du temps, de la stabilité et l'association des agents concernés. Elle s'est poursuivie néanmoins, en particulier au sein de l'administration de Bercy. L'un des principaux points d'achoppement reste la fiscalité environnementale

de l'équilibre financier des entreprises et de l'équité pour les ménages engagés dans cette transition énergétique. Autre point d'achoppement majeur : l'ajournement de la réforme des retraites du fait de la crise sanitaire. Si son opportunité pouvait faire débat en 2019, le retour de déficits importants dans l'ensemble des comptes de la sécurité sociale laisse imaginer quels efforts seront nécessaires quoi qu'on en dise pendant la prochaine campagne électorale. Il est néanmoins certain qu'une telle réforme ne pouvait être engagée par le biais d'un simple amendement au PLFSS.

moindre recours aux décrets d'avance, qui contournent l'autorisation parlementaire, limitation du PLFR de fin d'année à un texte de fin de gestion, travaux menés à l'Assemblée nationale

Sur le plan des dépenses, ce quinquennat aura été marqué par le renforcement des budgets régaliens, défense, intérieur, justice, mais aussi par un réinvestissement dans l'enseignement, sans oublier le système de santé, qui s'est retrouvé au coeur de la crise sanitaire.

dans le cadre de réformes telles que la loi Engagement et proximité. Je souhaite à ce stade évoquer les contraintes inhérentes au statut de parlementaire lors de l'examen des projets de loi, recevabilité financière définie par l'inflexible article 40 de la Constitution et règles anti-cavaliers. Ces dispositions limitant l'initiative parlementaire, qui découlent du parlementarisme rationalisé cher aux fondateurs de la V République, ne s'appliquent bien sûr pas au Gouvernement,

épidémique du covid-19. Je note toutefois que les nombreux dispositifs de soutien émanant de nos travées et de l'action gouvernementale ont bel et bien porté leurs fruits. Le taux de croissance devrait en effet dépasser cette année les 6 %. Il est inutile de se réjouir trop vite : nous nous trouvons dans une situation de rattrapage par rapport à 2020, et non dans un schéma de pleine reprise économique. Concernant le budget de l'année 2022,

de 13,4 milliards d'euros par rapport à la prévision révisée pour 2021, celles-ci s'établissant dès lors à 292 milliards d'euros. L'objectif est clair : le projet de budget pour 2022 a pour ambition d'illustrer, selon les mots du Gouvernement lui-même, une « normalisation progressive des finances publiques

après son annulation l'an dernier. Nous proposerons également des amendements d'aide aux associations, en reprenant la proposition de loi de notre collègue Éric Gold visant à encourager les dons et adhésions aux associations à vocation sportive et culturelle.

France dans le monde. J'ai relevé par ailleurs des mesures qui auront des conséquences importantes dans les domaines concernés : la poursuite de la reprise de la dette ferroviaire à hauteur de 10 milliards d'euros, l'expérimentation de la recentralisation du RSA dans les départements volontaires, les multiples mesures prises en faveur des professionnels indépendants ou encore la réforme par ordonnance du régime de responsabilité des comptables publics. Je conclurai mon intervention par une brève considération sur la période qui s'ouvre : nous savons bien qu'un budget préélectoral peut comporter des mesures exceptionnelles. Alors que les citoyens seront bientôt appelés à se prononcer dans le cadre du rendez-vous politique majeur de notre pays, mon groupe tient à rappeler son attachement au débat parlementaire dans sa plénitude : examiner

de ses voisins européens, une reprise de l'économie, mais il fait face aussi à un regain de l'épidémie. Or il est difficile de

La législature s'est ouverte sur la suppression de l'ISF et l'exécutif n'a cessé, depuis, de privilégier les entreprises et les plus riches de nos concitoyens : instauration de la sur les revenus du capital ; baisse des impôts de production pour les entreprises, même les plus prospères

qu'elle ait permis 1,1 milliard d'euros d'économies quand tant de Français modestes, de jeunes, de familles, vivent des situations très difficiles. Si la liste est longue, la finalité est toujours la même ce sont les catégories populaires et la classe moyenne qui doivent payer la facture, mais aussi les générations futures, l'accroissement du déficit et de la dette. Et ce sont les plus riches et les entreprises- même les plus grandes, même celles qui font le plus de bénéfices -qui sont préservés, pour des raisons idéologiques.

une politique injuste, douce avec les riches, mais dure avec ceux qui sont déjà le plus en difficulté, comme l'illustre la réforme de l'assurance chômage.

l'instant ! Les Français doivent se méfier de cette contradiction, qui relève soit du double discours soit de la navigation à vue. Le groupe socialiste n'a jamais cru à la théorie du ruissellement : en plus d'être inefficace, elle renforce les inégalités.

Pour ce qui est de l'absence de politique volontariste de redistribution, les différences entre la droite sénatoriale et le Gouvernement relèvent souvent de l'épaisseur du trait.

par ailleurs de la méthode du Gouvernement ? Que dire du plan France 2030, doté de 34 milliards d'euros en autorisations d'engagement et introduit par voie d'amendement à l'Assemblée nationale

Les parlementaires ne sont d'ailleurs pas les seuls à s'en offusquer puisque, pour la première fois, le Haut Conseil des finances publiques a refusé d'émettre un avis sur le volet dépenses

le sais bien, la période de précampagne présidentielle n'est pas pour rien dans cette situation. Personne n'est dupe : ces annonces s'apparentent davantage à de la communication et à du saupoudrage qu'à une réelle volonté de résoudre les problèmes auxquels le pays et nos concitoyens sont confrontés.

Les économistes de l'Institut des politiques publiques, disais-je, ont simulé l'effet des mesures fiscales et sociales mises en oeuvre pendant le quinquennat sur le niveau de vie des ménages. Mais, contrairement à la direction générale du Trésor, qui a classé les ménages par décile,

On retrouve le fil conducteur de la politique budgétaire et fiscale du Gouvernement : une injustice qui accroît les inégalités sans dynamiser la croissance. C'est l'échec du ruissellement Rien dans ce projet de budget pour 2022 ne vient malheureusement rectifier cette trajectoire. Nous ne saurions donc nous y reconnaître.

ce budget est également un budget sincère et cohérent, mais j'aurai l'occasion d'y revenir. Le PLF pour 2022 traduit la poursuite de la mise en oeuvre des engagements pris par le Président de la République depuis 2017 tout faire pour améliorer la compétitivité de notre économie et augmenter le pouvoir d'achat des Français. C'est la relance par la compétitivité qui nous permet de financer notre modèle de protection sociale et d'accompagner les plus vulnérables au coeur de la crise. Poursuivre la mise en oeuvre des engagements pris,

d'habitation sur les résidences principales, qui concernera enfin 100 % des Français en 2022. Des paroles aux actes, il y a parfois un long chemin. Depuis 2017, la majorité présidentielle, elle, aura tenu ses engagements. C'est le budget des promesses tenues, donc, mais aussi budget adapté et prudent en vue de la sortie de crise. La politique du « quoi qu'il en coûte » était nécessaire, mais elle a surtout été efficace ! Sans elle, combien de faillites inévitables aurait-on eu à déplorer ? Les mesures de soutien prises par le Gouvernement

conduit à rester prudents et à redéfinir un certain nombre de dispositifs. Les nouveaux scénarios de croissance et la réduction du déficit public, qui sera quasiment divisé par deux en 2022 et devrait atteindre un niveau inférieur à 5 %, apportent leur lot de bonnes nouvelles. serait toutefois dangereux d'arrêter brutalement les dispositifs de soutien en pleine phase de reprise et de laisser les entreprises face au mur de la dette. C'est pourquoi la date limite d'octroi des prêts garantis par l'État a été prolongée du 30 juin au 31 décembre 2021. Ce budget est inédit, également, compte tenu des défis auxquels nous devons faire face. Nous devons redresser nos finances publiques en résorbant le déficit, tout en accompagnant la reprise. Le défi est de taille ; là est toute l'ambition de ce budget, à la croisée des chemins entre la sortie de l'urgence et la préparation de l'avenir. Cette ambition passe par une redéfinition de de nos grandes priorités et devra tracer un chemin pour les dix années qui viennent, en commençant par une relance durable l'accélération de la transition écologique. Dans ce projet de budget, 1,5 milliard d'euros supplémentaires sont ainsi alloués au ministère de la transition écologique. Pour reprendre en main le destin de notre pays, le Président de la République s'est engagé à renforcer l'indépendance de la France dans de nombreux secteurs d'avenir comme l'hydrogène, l'aéronautique ou les biomédicaments. Je parle bien entendu du plan France 2030, doté de 34 milliards d'euros sur cinq ans, inscrits dans le présent

pour la deuxième année consécutive. C'est une hausse historique au service des justiciables et de ceux qui travaillent au quotidien à ce que la justice tous les gouvernements précédents y avaient renoncé. Ce PLF consacre une revalorisation historique du budget destiné à l'aide juridictionnelle, qui s'est accru de près de 30 % depuis 2016. Nous nous étions engagés à renforcer les moyens du régalien : l'engagement sera tenu. Relancer la France ne sera évidemment possible qu'avec le soutien des collectivités territoriales. Préservée grâce au soutien de l'État durant la crise sanitaire, la situation des finances locales s'améliore nettement en 2021. Malgré des disparités, chaque niveau de collectivité bénéfice en réalité d'une hausse

Que l'on ne vienne pas nous parler ensuite de promesses électorales ! Et pourtant, je n'oublie pas que les collectivités ont besoin d'un soutien fort et durable de l'État. Avec ce budget, l'engagement pris depuis 2017 est tenu. Ainsi les dotations de fonctionnement sont-elles stables pour la cinquième année consécutive. L'expérimentation d'une recentralisation du RSA permettra aux départements qui le souhaitent

horizontale, élaboré en collaboration avec les régions. Chacun, dans cette assemblée, porte une attention particulière à nos territoires et aux élus qui les font vivre au quotidien ; or, vous le constatez, mes chers collègues, les concours financiers de l'État aux collectivités territoriales progressent de 525 millions d'euros par rapport à 2021. À aucun moment nous ne nous sommes servis de la crise pour baisser les dotations. Bien au contraire, les collectivités se portent aujourd'hui mieux qu'en 2017 grâce à une augmentation de leurs investissements, de leur épargne brute et de leur trésorerie. Je n'oublie pas que nos élus locaux n'ont pas ménagé leurs efforts et méritent la confiance renouvelée que leur accorde l'État à travers ces moyens financiers de finances est un budget pour l'avenir des territoires. Le plan de relance ouvre notamment 1,2 milliard d'euros de crédits pour soutenir les actions en matière d'emploi ou d'infrastructures de transport fluvial et ferroviaire.

avec des droits et des devoirs ! Notre objectif est clair : aider au moins 400 000 jeunes en 2022. Certains qualifient ce projet de loi de finances d'électoraliste ; d'autres parlent d'un budget insincère, voire incohérent. Je compte répondre à ces accusations. L'insincérité, tout d'abord : il me semble que les mots ont un sens.

d'« insincérité » n'était pas approprié. Mes chers collègues, je l'affirme aujourd'hui à cette tribune : ce budget est complet, sincère et cohérent ! Mais Symbolise-t-il un chéquier illimité destiné à faire campagne ? Certains candidats n'ont pas manqué de créativité ou de mauvaise foi pour le dénoncer, souvent, d'ailleurs, de façon contradictoire. Peut-on, dans le même temps, parler d'une cagnotte constituée sur le dos des Français et dénoncer un budget qui ferait sauter toutes les digues et « cramerait la caisse » ? Je mets nos détracteurs au défi de nous proposer la suppression de l'une ou l'autre de ces mesures, ... Nous l'avons fait hier ! ... sans doute parce qu'au fond ils en approuvent chacune des composantes. Veulent-ils revenir sur l'augmentation de l'aide juridictionnelle ? Veulent-ils renoncer à l'augmentation des bourses sur critères sociaux, aux revalorisations décidées lors du Ségur de la santé ? J'observe du reste que ces mêmes responsables politiques ne refuseront

ce budget protège largement nos concitoyens, et c'est heureux, car les Français font aujourd'hui face à une situation alarmante en raison de l'inflation. Veuillez conclure. Le bouclier tarifaire voté pour contrer la hausse des prix de l'énergie, ce sont 5 milliards d'euros rendus au Français.

Les positions des uns et des autres répondent à des tactiques qui n'ont, au fond, pas grand-chose à voir avec la gestion des finances publiques. Si l'on adopte la seconde méthode, le projet de loi de finances pour 2022 révèle la politique menée depuis 2017. Il fait apparaître les succès et les échecs, les avancées et les lacunes. Bref, il permet de dresser un bilan de l'action gouvernementale. Pour ne rien vous cacher, monsieur le ministre, mes chers collègues, je crains que nous cédions cette année aux sirènes de la première méthode. Je tâcherai pour ma part, humblement, d'éviter cet écueil, mais je pense utile d'aborder d'emblée les critiques qui sont adressées à ce budget. On dit de ce projet de loi de finances pour 2022 qu'il est insincère et incomplet. Insincère, parce que les mesures qu'il contient ne répondraient qu'à des objectifs strictement électoraux. Incomplet, parce que le texte a été, depuis sa présentation en conseil des ministres, augmenté de nombreuses mesures, au gré des annonces de l'exécutif. Sur ce second point, si l'on préfère voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, on peut dire que le Gouvernement a complété le texte au fur et à mesure. Cette situation présente au moins un avantage pour le Sénat : nous aurons le loisir, pour ce qui nous concerne, de débattre d'un texte complet, du moins je l'espère.

À l'instar de nombreux collègues de la majorité sénatoriale, j'ai été rassuré de constater qu'il ne s'agissait pas, sous couvert d'un nouvel acronyme, d'un RSA jeunes. La mesure vise au contraire à renforcer la garantie jeunes, qui a fait ses preuves. meilleure manière de l'articuler avec les dispositifs existants. Ainsi présenté, ce contrat d'engagement semble cibler les publics les plus éloignés du marché de l'emploi, ceux-là mêmes qui ne bénéficient pas de l'amélioration du marché du travail. également susceptible de simplifier le panel des solutions proposées aux jeunes. Il offre donc davantage de lisibilité et de clarté aux acteurs de terrain. Cependant, le Sénat, dans sa grande diversité, demeure très attaché au rôle que jouent les missions locales dans le maillage des politiques d'insertion des jeunes. À cet égard, monsieur le ministre, force est de constater que la lente incubation du dispositif dans les arcanes de Bercy, puis sa précipitation brutale dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale n'ont pas permis d'atténuer toutes les inquiétudes. J'espère que nous aurons l'occasion d'en débattre : c'est ainsi que nous pourrons faire entendre la voix des élus dans l'élaboration de ce budget. Pour ce qui concerne le premier point, à savoir la prétendue insincérité du budget, nos débats, là encore, devraient permettre de lever les doutes sur certaines des interrogations légitimes qui ont été formulées.

Or nous nous trouvons aujourd'hui dans une conjoncture des plus paradoxales. D'une part, la reprise économique est forte. Les bons résultats valident la stratégie, adoptée par le Gouvernement et approuvée par le Parlement, de soutien aux entreprises et aux ménages.

D'autre part, l'épidémie menace de reprendre partout dans le monde, en Europe plus vigoureusement qu'ailleurs. En Allemagne, justement, l'augmentation fulgurante du nombre de cas incite à la plus grande vigilance sanitaire. Surtout, cette instabilité chronique nous oblige à naviguer à vue en matière économique, car les indicateurs conjoncturels ne valent désormais plus que pour quelques mois, si ce n'est pour quelques semaines. Pour ne pas nous égarer, nous devons nous en remettre à notre boussole. Il s'agit de combiner le court terme et le long terme, d'articuler la tactique et la stratégie, de parer à l'urgence présente, tout en préparant l'avenir.

ménages bénéficient d'une revalorisation du barème de l'impôt sur le revenu destinée à neutraliser les effets de l'inflation, ainsi que de la suppression de la taxe d'habitation pour tous les Français. Pour les entreprises, le Gouvernement propose de maintenir la trajectoire de baisse de l'impôt sur les sociétés et des impôts de production. Ces mesures doivent nous permettre d'accélérer la réindustrialisation de notre pays et de conserver les centres de décision en France, en évitant de futures délocalisations. Elles font même dire à certains élus de gauche qu'il s'agit d'un budget de droite Le message envoyé est clair : la France valorise mieux le travail. Les efforts de nos concitoyens paient mieux. Leur niveau de vie s'améliore, et l'État les protège en cas de coup dur. Cette stratégie du Gouvernement a de quoi rassurer tous les tenants d'un gaullisme social fondé sur la promotion du travail. Dans cette logique, je tiens aussi à insister sur les diverses mesures qui déclinent, au niveau fiscal, le plan Indépendants. Celles-ci visent à compléter le projet de loi que nous avons adopté le mois dernier, et qui permettra de simplifier la vie de tous les indépendants, de tous les commerçants, de tous les artisans, de tous les libéraux, bref, de tous ceux qui, en France, se font une certaine idée de l'autonomie et du travail. Nous ferons plusieurs propositions pour amplifier la portée de ces mesures et soutenir ces hommes et ces femmes ; ils ont tenu bon pendant la crise et ne doivent pas être les grands oubliés de la reprise. C'est une question de justice fiscale, c'est-à-dire de répartition équitable des contributions selon les efforts et les mérites. La justice fiscale ne saurait se réduire à une formule toute faite, que l'on utiliserait à l'envi pour taxer davantage les Français.

La politique fiscale du Gouvernement, qui a allégé le fardeau fiscal qui pesait sur les ménages et sur les entreprises, ne doit pas se faire aux dépens des collectivités locales. Notre groupe accueille donc favorablement la proposition

en consolidant les crédits des armées, de la justice et de la police. Depuis 2017, nous affirmons notre attachement à cet engagement, et nous persistons dans cette voie. La commission des finances ne s'y est d'ailleurs pas trompée en adoptant les crédits de chacune de ces missions régaliennes. Ce faisant, nous nous donnons les moyens de remettre de l'ordre dans notre pays. C'est ce qu'attendent les Français, mais ces efforts ... Veuillez conclure. ... ne doivent pas se faire au détriment de notre souveraineté économique. C'est pourquoi il nous faudra, sans tarder, remettre de l'ordre dans nos finances publiques.

Merci, madame la présidente ! Il n'aura échappé à personne que ce budget est le dernier du quinquennat.

Nous déplorons qu'aucune mesure d'économie ne permette de compenser ces dépenses. Toutes les réformes ambitieuses du quinquennat en matière d'économie ont été abandonnées- je pense à la réforme des retraites ou à la diminution du nombre de fonctionnaires -, et ce avant même le déclenchement de la crise. Dépenser n'est pas réformer ! Depuis 2015, la France est la championne des dépenses publiques au sein de l'OCDE. Le « quoi qu'il en coûte » perdure même après la crise : catégorie de population après catégorie de population, des chèques en bois sont signés de nombreuses dépenses nouvelles sont pérennes ou engagées sur plusieurs années : elles pèseront sur les budgets du prochain quinquennat, obérant la capacité du prochain Président de la République à redresser les comptes publics. Quelle que soit la légitimité des besoins, la multiplication des chèques quelques mois avant l'élection présidentielle, personne n'est dupe de la finalité électoraliste de telles mesures. Si la crise a détérioré de manière exceptionnelle nos finances publiques, elle a aussi mis en lumière nos faiblesses et l'absence d'efforts antérieurs.

Conséquence de ces déficits considérables : notre dette publique est bien plus importante que celle des États voisins. Comme l'a très bien dit le gouverneur de la Banque de France, notre problème

Au regard de l'ensemble de ces indicateurs, crise ou pas crise, ce quinquennat aura été un échec. La France, initialement moteur de l'Europe avec l'Allemagne, est aujourd'hui un frein au redressement de l'économie européenne

Par ailleurs, des décisions de justice récentes condamnent l'État pour inaction. Le tribunal administratif de Paris lui a imposé récemment de réparer les conséquences de sa carence en matière de lutte contre le réchauffement climatique. Selon les juges, et malgré l'aide de la covid-19, les engagements fixés dans la stratégie nationale bas-carbone pour la période 2015-2018 sont atteints à 15 millions de tonnes équivalent CO2 près. Par arrêt du 15 novembre 2021- c'était cette semaine -, le Conseil d'État ordonne au Gouvernement d'agir pour réduire de façon draconienne l'utilisation des pesticides dans les sites Natura 2000.

Je remarque d'ailleurs avec malice que cette politique ne va pas dans le sens de l'émancipation par le travail prônée par le candidat-président. Vous créez également un sentiment d'inquiétude dans les milieux économiques. Interrogé sur France Info, Geoffroy Roux de Bézieux a qualifié a qualifié l'indemnité inflation de « dangereuse » car elle « met dans la tête des Français l'idée qu'on va compenser systématiquement l'inflation par des mesures d'aides gouvernementales. Cela ne peut pas marcher.

Par ailleurs, certaines pratiques, dérogatoires au principe d'universalité budgétaire, sont peu compatibles avec l'autorisation parlementaire des dépenses de l'État. Je ne prendrai qu'un exemple, du programme 204. En 2020, pas moins de 700 millions d'euros issus d'un fonds de concours alimenté par des versements de Santé publique France, agence désormais financée intégralement par l'assurance maladie et dont la et dont la dotation échappe au contrôle parlementaire, ont été rattachés à ce programme. Le détail des dépenses du fonds de concours n'est retracé nulle part dans les documents budgétaires, alors même que celles-ci ont représenté plus du triple des crédits ouverts sur le programme en loi de finances initiale pour 2020. Le présent projet de loi de finances, tout comme le PLF pour 2021, ne remet pas en cause cette architecture.

dont plus de 20 prorogations, renforcements ou créations de niches fiscales- autant de pertes de recettes non chiffrées qui auront un impact sur le prochain quinquennat. Mais ce sont

11,8 milliards d'euros de dépenses ont été ajoutés à l'Assemblée nationale. Qu'en serait-il à la sortie du Sénat, puisque les quarante annonces des trois derniers mois représentent 25 milliards d'euros de dépenses supplémentaires pour 2022 et 65 milliards d'euros sur le prochain quinquennat ? cet égard que certaines promesses, notamment celles qui ont été faites aux personnes âgées en perte d'autonomie et pour le développement du fret ferroviaire, le remboursement des consultations chez les psychologues ou l'élargissement du Pass'Sport, n'ont toujours pas de traduction budgétaire.

». Pour plus de facilité, ou peut-être pour cause d'impréparation, le plan France 2030 a été intégré dans la mission « Investissements d'avenir ». La Cour des comptes, dans un référé de juillet 2021, n'a pourtant pas manqué d'émettre

entre les programmes de la mission « Investissements d'avenir » est qualifiée de « première ébauche », la répartition pouvant évoluer « en fonction de la réussite des dispositifs sous-jacents

une partie du prix du mégawattheure est, elle, indexée sur le prix du gaz, en lien direct avec la croissance des énergies renouvelables intermittentes dans le mix électrique. Qu'en sera-t-il cet hiver si, malheureusement, il n'y a pas de vent ? La France a maintenant besoin de mesures pérennes et structurelles pour garder une indépendance et une souveraineté énergétiques à des prix corrects pour les Français et leurs entreprises. Or le soutien à la filière hydrogène et au nucléaire relève encore trop de l'effet d'annonce. Alors que 600 millions d'euros devaient être consacrés à la production

Le plan de relance consacre seulement 200 millions d'euros à la filière nucléaire ; quant au plan France 2030, il lui alloue 1 milliard d'euros d'ici à 2030. Le prochain gouvernement ne devra pas enjamber le passage devant le Parlement à l'occasion de la révision de la PPE. Autre défi, la fiscalité locale. Les effets de la suppression de la taxe d'habitation et d'une partie des impôts de production sur les indicateurs synthétiques auxquels est adossé le système des finances locales, et le lissage de ces constituent une véritable bombe à retardement pour les mécanismes de péréquation, déjà minés par l'obsolescence des indicateurs. Avec la révision des valeurs locatives en 2026, les élus ne disposent plus d'aucune lisibilité sur leurs finances. Ils anticipent, après les échéances du printemps, un tour de vis sur les dotations de l'État pour faire face au mur de la dette. Ce contexte

Par un tour de passe-passe, celle-ci évolue de 115 % à 114 % du PIB entre 2021 et 2022. Or le déficit sera de l'ordre de 125 milliards d'euros

pourrait conduire notre pays à la catastrophe. Le remboursement de la dette ne peut reposer que sur une croissance corrélée à la maîtrise, à défaut d'une baisse, de la dépense publique. Le PLFR que nous avons examiné hier et, plus encore, le PLF dont nous allons débattre au cours des prochains jours ne suivent absolument pas cette voie. Il nous incombe d'être responsables à l'égard des Français, notamment des générations futures. Le groupe Les Républicains refuse le chemin de la facilité et de la démagogie. Nous ne voterons donc pas ce texte, par respect pour les Français.

ce projet de loi de finances nous parvient dans un contexte que nous espérons toutes et tous être un contexte de sortie de crise : la croissance est là, mais elle ne peut masquer un nombre important de besoins sociaux et environnementaux non satisfaits.

d'une récente étude, sur laquelle s'appuie le Gouvernement, prétendent que le taux de pauvreté serait stable, à un niveau tout de même très élevé de 15 %. Mais sont exclus de l'échantillon beaucoup d'étudiants, de personnes sans domicile fixe et de personnes travaillant dans le secteur informel, c'est-à-dire de personnes très très exposées à la pauvreté. Il est donc fort probable que le taux de pauvreté ait en réalité augmenté. Les associations de solidarité le vivent au quotidien. Nous ne saurions négliger le fait que 20 % des Français ont froid chez eux l'hiver, ou encore que 20 % d'entre eux déclarent sauter certains repas

monsieur le ministre : les inégalités progressent et votre politique fiscale n'a fait qu'amplifier ce phénomène. Les classes moyennes sont par ailleurs touchées par un retrait majeur du service public dans les territoires. Face à cette situation, que fait le Gouvernement ? Il mène une politique fondée sur l'offre, un plan de relance et un plan d'investissement qui sont avant tout des plans de subventions aux entreprises sans conditionnalité, ne portant ni objectif stratégique ni véritable ambition de transformation verte.

La politique consistant à clamer haut et fort que le chômage diminue, que tout va bien, que de très nombreux emplois ne sont pas pourvus est une vaste supercherie. Elle sert à justifier le discours de culpabilisation des chômeurs, qui lui-même sert à justifier la baisse des dépenses publiques au détriment de leurs indemnisations, et ce pour financer les baisses d'impôts

Quant aux mesures environnementales et climatiques, elles sont très insuffisantes face à une situation que tout le monde qualifie pourtant de situation d'extrême urgence. Sécheresses, incendies, inondations, canicule : tout le monde est touché ; la France aussi, bien entendu.

si cette amélioration est par ailleurs insuffisante pour respecter les engagements internationaux de la France. Par conséquent, ce budget vert est inopérant. Dans sa nouvelle version, le nucléaire est par ailleurs classé comme énergie totalement propre,

Pendant ce temps, en raison de la fraude fiscale, la France perd chaque année 17 milliards d'euros de recettes d'impôt sur les sociétés, soit 40 % des recettes de cet impôt. L'évasion fiscale permet aux 1 % les plus riches de réduire leurs impôts sur le revenu d'un montant pouvant atteindre 30 % des impôts dus.

vous avez sciemment laissé faire et vous vous obstinez dans ce choix, en poursuivant la restriction des effectifs dans les services de contrôle fiscal. Ainsi, au terme de ces cinq années de présidence, on voit bien que ce quinquennat est celui des inégalités et qu'Emmanuel Macron est le président des riches. Au moment de la suppression de l'ISF, vous aviez promis de revoir votre copie si cette politique s'avérait inefficace. Elle l'est, tout le monde le dit et les rapports le montrent

de budget, on le voit, ne répond pas aux grands enjeux : réduire les inégalités, affronter le dérèglement climatique. Mais je voudrais prendre quelques instants pour évoquer la méthode employée. On a le sentiment, depuis le mois de septembre, que le Gouvernement a le carnet de chèques bien ouvert.

Mais les largesses d'aujourd'hui sont financées par l'austérité de demain, que vous vous proposez de mettre en oeuvre en cas de réélection, comme vous l'avez écrit à la Commission européenne en avril dernier, dans le cadre du programme de stabilité. Loin d'utiliser le poids de la France pour faire de la sortie de crise un moment fort de rupture avec la logique d'austérité des traités européens, vous confortez cette logique et vous engagez, pour le prochain quinquennat, à revenir sous le seuil des 3 % dès 2027, une trajectoire de limitation de l'augmentation des dépenses

Au vu de l'angoisse climatique qui se développe au sein de notre jeunesse, après des mois d'une crise très dure qui l'a mise en danger, il faudrait une vaste politique permettant à chaque jeune de trouver sa voie, de construire sa vie et son projet, afin que toute notre société bénéficie de ses potentialités.

il fallait travailler à offrir de réelles chances à notre jeunesse. Mais, même aux étudiants qui réussissent, vous n'offrez aucune perspective ; vous êtes incapables de leur permettre ne serait-ce que de poursuivre leurs études- je pense ici à ces milliers de jeunes qui ont obtenu leur licence avec de bons résultats et qui, n'ayant pas de master, master, sont obligés de s'exiler en Belgique, dans le meilleur des cas, pour avoir une chance de continuer leur cursus. Je pense aussi à tous ces jeunes broyés par cet abominable logiciel Parcoursup, qui crée de l'angoisse chez les élèves dès la première et les trie sans aucun égard pour leurs rêves, leurs souhaits, leur avenir. Et je pense à ces jeunes qui, en lycée professionnel, ont vu baisser leurs heures d'enseignement général, au mépris de la formation de citoyen à laquelle ils ont droit. Ce projet de budget n'est décidément par pour elles ni pour eux, qui pensent à l'avenir, qui n'osent pas espérer, mais qui attendaient à tout le moins de la France qu'elle soit à la hauteur des enjeux à Glasgow. Cette jeunesse vaut mieux que des concours d'anecdotes, et vous la méprisez par une politique qui insulte l'avenir

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, notre question préalable ne valait pas fermeture au débat, mais appel à un vote sanction- sanction d'un budget toujours plus discriminant et béotien. Nous ferons, amendement après amendement, proposition après proposition, la démonstration de l'échec de ce quinquennat.

Restaurer les finances publiques ? Vous avez réduit d'au moins 52 milliards d'euros les recettes de l'État de façon pérenne. Retrouver le chemin de la croissance ? L'activité avait reculé de 18 % au second trimestre de 2020, soit un quart de plus que la moyenne européenne. Baisser le chômage ? Depuis le début du quinquennat, il y a tout de même 17 000 demandeurs d'emploi supplémentaires. Augmenter le pouvoir d'achat ? Les plus riches ont bénéficié de 3 518 euros en moyenne ; les plus modestes ont encore perdu 35 euros par an. Restaurer la « compétitivité » de l'économie française ? Le solde de la balance commerciale est négatif de 60 milliards d'euros en moyenne sur le quinquennat, attestant la dépendance de la France aux importations étrangères. On le sait, « l'éloge des absents se fait sans flatterie ». Le ministre Bruno Le Maire avait tort le 31 mai 2021 ; il a tort en novembre 2021 ; il aura probablement tort en 2022. Non, les indicateurs économiques ne sont pas bons

Vous avez commencé par détricoter le code du travail, en légitimant le plafonnement des indemnités de licenciement et en consacrant les accords d'entreprise au détriment des accords de branche. sauront qui les a privés de leurs droits face au patronat. Peu après, dans le cadre du projet de loi de finances pour 2018, vous avez supprimé l'impôt de solidarité sur la fortune et restauré l'. Pourtant, aucun ruissellement n'a coulé sur l'économie réelle. L'année suivante, la loi portant a impulsé une véritable dynamique, celle du démantèlement des financements publics de l'habitat social. Le secteur privé a gagné le droit de construire plus vite, moins bien et plus cher.

pension. C'est à cette même période qu'apparaît le chèque énergie, remplaçant les tarifs sociaux de l'énergie et matérialisant l'incapacité du Gouvernement à anticiper la hausse de la facture pour nos concitoyens. Nous ne sommes qu'en mai 2019 lorsque le démantèlement de l'État se traduit dans la loi Pacte, ce même État détenant 124 milliards d'euros de participation dans des entreprises stratégiques, sans compter le capital détenu par la Banque publique d'investissement, laquelle n'est pas, nous dit-on, un « bon actionnaire » -. Il vous a fallu privatiser la Française des jeux,

qui, une fois la crise sanitaire arrivée, n'ont pu ignorer la SNCF, EDF ou Air France-KLM, comme si l'État avait finalement une raison d'être dans ces secteurs. Vient ensuite cette « taxe vitrine » sur les géants du numérique,

Madame la présidente, monsieur le ministre- merci de votre présence constante et attentive à nos côtés

D'un point de vue économique, le choc de la crise du covid-19 a été largement absorbé par les finances publiques. Si nous n'en remettons pas en cause le bien-fondé stratégique, le « quoi qu'il en coûte » a un prix : la dette. Et l'État providence a ses limites, temporelles et structurelles. La limite temporelle sera vraisemblablement atteinte dans douze mois, avec la fin probable de la clause dérogatoire générale du pacte de stabilité et de croissance La limite structurelle, quant à elle, a été franchie avant même la pandémie, la dette publique ayant dépassé le seuil symbolique de 100 % du PIB en septembre 2019. Désormais tournés vers la sortie de crise et contemplant nos comptes publics plus éprouvés encore qu'auparavant, nous pouvons nous réjouir que la charge de la dette reste faible. C'est justement parce qu'elle l'est, et parce que la croissance repart avec force, que notre groupe estime que la priorité budgétaire doit être donnée à la vertu. Lorsque les taux d'intérêt finiront par remonter, il sera trop tard. Dans le cadre de l'examen du projet de loi de finances pour 2022, le groupe Union Centriste portera une parole de responsabilité budgétaire globale. À cet effet, nous défendrons par voie d'amendement des dispositions visant à assainir nos finances publiques, tantôt à travers des recettes fiscales supplémentaires tantôt à travers des mesures d'économies budgétaires, autant de pistes permettant d'affecter davantage de moyens au service de la dette.

L'Observatoire français des conjonctures économiques, dans une note d'avril dernier, précise qu'une consommation d'un cinquième de cette épargne conduirait à une croissance du PIB de 2 points supplémentaires. Orienter davantage l'épargne vers les fonds propres de nos entreprises constituerait véritablement un puissant moteur pour notre activité économique et notre souveraineté nationale, sans recours à la dépense publique.

Mais il nous importe que les Français restent souverains et que, l'épargne nationale, ils détiennent le patrimoine national industriel ou stratégique, quel qu'il soit.

Face à la menace persistante d'une inflation prolongée, face à une pénurie de main-d'oeuvre et de matières premières qui s'annonce durable, nous ne pouvons que nous interroger sur la pertinence du lancement du plan France 2030 dès l'année 2022. À force de milliards, notre économie s'expose paradoxalement à la surchauffe. Il nous paraît plus cohérent de nous attacher dans un premier temps à concentrer l'effort public sur la consommation des programmes d'investissements d'avenir existants et du reliquat de 30 milliards d'euros de France Relance.

Notre filière bois, comme le secteur de la construction dans son ensemble, est fragilisée par la forte hausse du coût des matières premières. Ce phénomène conjoncturel, qui s'ajoute à une fragilité structurelle en capital, aggrave la situation de nos entreprises sur ce marché très concurrentiel à l'international. La place de l'État est à leurs côtés. Enfin, un budget ne saurait être vertueux sans donner à notre administration les moyens de lutter contre les fraudes fiscale et sociale.

du ministère de l'économie et des finances, afin qu'il puisse continuer à remplir ses missions en la matière. Le temps du retour à la normale implique une vigilance particulière quant à nos comptes publics.

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, « mieux vaut un raccommodage qu'un trou ». Cette maxime résume à elle seule tous les écueils du budget qui nous est proposé.

une seule a été choisie : les autres ont été dictées par un agenda sur lequel le maître des horloges n'a eu aucune prise. Nul doute qu'aujourd'hui, sans ces événements, la première période aurait été la seule : il se serait agi, Pourtant, entre le mouvement des gilets jaunes et la crise sanitaire, nous aurions pu imaginer une autre voie que celle qui fut ouverte au début du quinquennat. Force est de le constater : tel n'a pas été et tel ne sera pas le cas. Les très riches restent les grands gagnants des choix fiscaux de votre gouvernement. Selon une évaluation de l'Institut des politiques publiques, entre 2017 et 2022, les mesures sociales et fiscales ont fait augmenter de 2,8 % le niveau de vie du 1 % des Français les plus aisés, qui- je le rappelle -vivent avec 126 654 euros en moyenne par an, soit un gain moyen de 3 518 euros. En même temps », le niveau de vie du 1 % le plus pauvre a baissé de 0,17 %, soit une perte de 9 euros sur le quinquennat. Il semblerait que la boussole politique ait pour nord les premiers de cordée ; tant pis si même Joe Biden nous explique que le ruissellement est une fable. L'important, c'est que notre Président y croie vraiment : cela conforte sa foi dans le bien-fondé de ses mesures. mesures. Le million de pauvres supplémentaire qui découle de la crise sanitaire est souvent cité. Derrière ces données, il y a des femmes et des hommes à qui, à peine arrivés au pouvoir, vous avez commencé par supprimer 5 euros d'APL, avant de les trahir, au coeur de la crise sanitaire, en refusant d'augmenter les minima sociaux ou de les étendre aux moins de 25 ans. Vos politiques n'ont eu aucun effet sur l'investissement. Personne n'est surpris, si ce n'est vous, qui feignez de l'être. Le fait était prévu, d'ailleurs. Il a également été confirmé par les études que le Gouvernement a commandées à France Stratégie celles-ci concluent à l'impossibilité d'établir un lien entre les réformes de la fiscalité du capital et un accroissement des investissements ou des créations d'emplois. Affirmer le contraire- vous le faites régulièrement -relève au mieux de la naïveté, au pire du mensonge. Mais je ne m'étendrai pas davantage sur cet inventaire : mon collègue Rémi Féraud a déjà eu l'occasion de l'aborder. Concentrons-nous sur ce budget. Le PLF 2022, comme le PLFSS récemment adopté, ne comporte aucune mesure notable en ce qui concerne les ressources publiques, impôts ou cotisations sociales. Toutefois, la baisse de l'impôt sur les sociétés se poursuit, pour 3 milliards d'euros. La baisse de la taxe d'habitation rapportera 2,8 milliards d'euros aux 20 % de ménages les plus aisés, lesquels bénéficieront de la même somme de 2,8 milliards d'euros je déplore la pratique récurrente consistant à autoriser les entreprises à verser des suppléments de rémunération défiscalisés et désocialisés. Le quinquennat Macron rivalise d'ingéniosité en la matière. seulement à la fameuse prime exceptionnelle de 1 000 euros que les entreprises peuvent verser à leurs salariés, mais aussi à votre lumineuse idée d'exonérer d'impôts et de cotisations sociales les pourboires des hôtels, cafés et restaurants versés par carte bancaire. Je le dis sans ambages : cette mesure incitera les entreprises à instaurer un pourboire quasi obligatoire de 20 %, comme cela se fait aux États-Unis, et à baisser en contrepartie les salaires fixes. Tous les salariés ont droit à des salaires garantis. j'estime que toutes les rémunérations doivent supporter les impôts et les cotisations sociales, non par dogme politique, mais parce que ces dernières ouvrent des droits aux prestations chômage et retraite. En cela, la désocialisation ou défiscalisation des salaires est un piège grossier, qui, de surcroît, se referme toujours sur les mêmes.

Néanmoins, il marque un tournant vers un capitalisme technologique vert, par lequel, sous couvert d'écologie, l'État finance les efforts d'adaptation des entreprises françaises. D'un côté, il peut être utile de financer certaines innovations vertes et d'aider les entreprises à produire en France. De l'autre, le concept de « capitalisme vert » est un oxymore. but des entreprises reste la maximisation des profits plutôt que le bien-être social. Leur gouvernance n'est jamais remise en cause et l'objectif de sobriété, que visaient la plupart des 149 mesures de la Convention citoyenne pour le climat, est oublié. De toute évidence, et malgré la crise sanitaire, il manque une réflexion d'ensemble sur l'évolution à long terme de l'économie française : quelle souveraineté économique voulons-nous ? Quel tournant écologique ? Quel plein-emploi ?

Ce dispositif est ouvert à tous les propriétaires, quels que soient leurs revenus, qu'ils soient occupants ou bailleurs, pour une somme totale annoncée de 2 milliards d'euros en 2022. Au regard du format retenu, je crains un fort effet d'aubaine : les propriétaires les plus aisés, ayant de toute façon prévu des chantiers de rénovation, pourront profiter de la prime pour effectuer ces travaux à moindre coût aux frais du contribuable. Vous ne cessez de vous présenter en chantres de la défense du pouvoir d'achat. Pourtant, les chiffres nous disent le contraire. Selon les statistiques publiées par le Trésor, le pouvoir d'achat augmenterait de 8 % entre 2017 et 2022. ce chiffre, que vous mettez en avant à la moindre occasion, ne prend pas en compte l'évolution démographique. Ainsi, le pouvoir d'achat aurait en fait progressé de 1 % par an, soit un gain annuel moyen de 334 euros pour une personne seule. D'ailleurs, les Français ne s'y trompent pas

Nous mesurons, bien sûr, l'impact de la crise sanitaire sur la vie de nos concitoyens, de nos entreprises et de nos collectivités territoriales. Et nous saluons le retour de la croissance et de la création d'emplois. Mais comment expliquer que la confiance dans l'action publique, entamée il est vrai depuis plusieurs décennies, Les Françaises et les Français sont lucides. Ils savent par expérience que les engagements sont rarement tenus et qu'un jour il faudra collectivement régler l'addition. Ils savent que l'argent facile, l'argent magique, l'argent gratuit n'existent pas.

réduction de 120 000 postes de fonctionnaires, dont 70 000 dans les collectivités territoriales, ce qui trahissait d'ailleurs d'emblée une volonté d'ingérence dans les exécutifs locaux. Sur tous ces points, bilan rime avec néant.

En mars dernier, le Premier ministre a confié à un groupe d'experts conduits par Jean Arthuis, garant de l'orthodoxie budgétaire s'il en est, le soin d'analyser la situation et de faire des propositions. Parmi celles-ci figurent la création d'une norme de dépenses pluriannuelle déclinée dans toutes les administrations publiques et la création d'un compteur des écarts, que l'Allemagne, l'Autriche et la Suède ont déjà mis en oeuvre. L'ensemble serait contrôlé par une institution budgétaire indépendante issue de la transformation du Haut Conseil des finances publiques. Après lecture approfondie du travail de Jean Arthuis, le Premier ministre a déclaré : « Ce rapport alimentera les travaux du Gouvernement sur la stratégie politique budgétaire post-crise, ainsi que les réflexions en cours avec le Parlement »,

En conclusion, et pour revenir à des considérations plus immédiates concernant ce projet de loi de finances, nous sommes satisfaits de voir exaucer certains de nos voeux, exprimés de longue date. Je pense notamment aux différents rapports consacrés aux transports et à la mobilité, à la transition écologique et au numérique, pour ne retenir que les sujets relevant de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable.

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, le Gouvernement se félicite d'avoir « stabilisé » les dotations des collectivités territoriales depuis 2017, après des années de réduction. vous-même ne résiste pas à l'analyse de ce PLF, le dernier d'un quinquennat marqué par une défiance inégalée entre le Président de la République et les élus locaux. Les conclusions du Congrès des maires, cet après-midi, ne suffiront sans doute pas à renouer avec des élus qui se sentent méprisés, isolés, abandonnés. Les communes ont perdu un impôt historique- la taxe d'habitation -, dont la dernière tranche disparaît avec ce PLF. Elles ont également perdu la moitié des impôts de production. Les départements, après les régions, doivent renoncer à leur dernier pouvoir de taux. Les compensations sont incomplètes et illisibles- ainsi du coefficient correcteur. Le paysage des finances locales n'a plus rien de cohérent et plus personne n'y comprend rien Le lien, décisif pour la cohésion sociale, entre les citoyens et leurs communes, départements et régions, entre les activités économiques et les collectivités territoriales, se distend. L'autonomie financière des collectivités, indispensable au respect du principe constitutionnel de libre administration, se réduit encore ; et cette recentralisation ne se traduit aucunement par un renforcement de la présence de l'État dans nos territoires, au contraire. la disparition de plus de 500 trésoreries depuis 2013. Or, moins l'État est présent, plus il se fait tatillon, exigeant et technocrate, à l'égard des communes notamment. Le recul des services publics se répercute sur les collectivités. Celles-ci doivent par exemple contribuer au financement des maisons France Service pour garantir une présence minimale de la puissance publique, ou encore prendre des initiatives face à la désertification médicale. L'efficacité économique n'est pas non plus au rendez-vous. Ce sont d'abord les plus grandes entreprises, celles qui en ont finalement le moins besoin, qui bénéficient de la diminution des impôts de production. Pour elles, le gain moyen est de plus de 9 millions d'euros, contre 940 euros seulement pour les très poursuit le mouvement de regroupement et de fusion des collectivités, malgré le mécontentement que suscitent les intercommunalités et les régions XXL. Les communes qui fusionnent sont davantage subventionnées, au détriment de celles qui veulent continuer à assurer la proximité et à faire vivre l'institution préférée des Français. Vous poursuivez la mise en concurrence entre collectivités. À enveloppes constantes, quand les dotations augmentent pour certaines, elles diminuent pour d'autres, à l'image de la DGF, qui a baissé pour plus de la moitié des communes en 2021. Nous défendrons d'ailleurs des amendements tendant à revaloriser la DGF en prenant pour base l'année 2013 et en tenant compte de l'inflation actuelle. Nous proposons aussi que l'augmentation de la dotation de solidarité urbaine (DSU) et de la dotation de solidarité rurale (DSR) ne se fasse pas au détriment des communes qui n'en bénéficient pas.

durant la crise sanitaire est sans commune mesure avec l'aide apportée à la sphère privée. Les collectivités ont pourtant été et restent en première ligne face à l'épidémie. La clause de sauvegarde devait apporter 750 millions d'euros à environ 12 000 communes. Or seules un peu plus de 3 600 d'entre elles seront concernées, pour 177 millions d'euros mobilisés. Nous proposons de redonner des moyens d'action aux collectivités, par exemple en compensant les mesures salariales concernant les agents de catégorie C, qui représentent l'essentiel de leur masse salariale. de leur masse salariale. En investissant, en prenant soin de nos concitoyens, les collectivités prennent part à la relance. Elles doivent être soutenues en ce sens ! Très bien

à une entreprise indienne pour qu'elle s'installe en France sur un marché très concurrentiel et saturé, mettant en péril un fleuron de notre industrie. Je ne suis pas sûr que la théorie suivie soit logique

Nous pouvons nous interroger sur la performance du modèle adopté, notamment par rapport aux pays comparables de l'Union européenne. Je vous rappelle qu'en 2020 l'Allemagne n'était qu'à 4,7 % de déficit quand nous étions à 9,1 % et que sa dette, au sommet de la crise, s'est élevée à 68,7 % de son PIB, contre 115

sur l'emploi de l'argent et sur ses effets. À aucun moment n'ont été proposés une politique sérieuse et un travail de concertation avec le Parlement pour rembourser la dette et relancer l'économie. Jamais nous ne nous sommes interrogés sur nos capacités à emprunter et sur les dispositifs à adopter pour rembourser. Cette gestion est irresponsable. Mais la gestion calamiteuse des finances de l'État ne trouve pas uniquement sa source dans la crise que nous venons de traverser. En réalité, votre gouvernement a la dépense facile et met aisément sur le dos du covid-19 les dépenses très politiques qu'il souhaite engager. J'en veux pour preuve que, depuis juillet 2021, alors que l'épidémie était au plus bas, le Président de la République a engagé pas moins de 25 milliards d'euros de dépenses supplémentaires. C'est insupportable ! Croyez-moi, les Français le pensent et s'en inquiètent.

Aucun des engagements formulés en matière de responsabilité financière par le Président de la République dans son programme de 2017 ne semble avoir été honoré. Au terme du quinquennat, la France est toujours championne d'Europe des dépenses publiques, toujours championne d'Europe des prélèvements obligatoires,

Vous avez souvent laissé planer l'idée que la gestion de l'État n'était pas à comparer avec celle d'un ménage ou d'une entreprise. Si tel est le cas, expliquez-moi alors pourquoi l'Allemagne ne suit pas votre théorie ! Comme notre dette propre ne vous suffisait visiblement plus, nous avons engagé un processus d'émission de dette commune avec les autres États membres de l'Union européenne- cette dette n'entre pas dans le calcul de la dette nationale, mais elle devra être remboursée par nos finances si nous n'arrivons pas à mettre en place des recettes européennes. C'est encore irresponsable

Aujourd'hui, l'épargne est une garantie ; mais si, un jour, vous ou votre successeur étiez amené à prélever sur l'épargne des Français, je pense que la confiance serait définitivement rompue et que l'épisode de gilets jaunes que nous connaîtrions serait autrement plus grave que celui que nous avons vécu. vécu. Au vu du chemin que nous empruntons- 45 000 euros pèsent sur la tête de chaque Français -, il est impératif de faire des choix courageux. De tels choix sont malheureusement absents de votre budget

Je n'ai toujours pas eu de réponse à ma question. Enfin, concernant les charges, vous adoptez la politique de la taxe plutôt que celle de la réforme d'un système devenu obèse et qui coûte trop cher. En réalité, vous préférez augmenter les recettes plutôt que réduire les dépenses, qui s'élèvent aujourd'hui à 57 % du PIB.

que toute dette est forcément négative, mais elle doit être une bonne dette, une dette d'investissement pour les générations futures, et rien d'autre. Or, aujourd'hui, la dette est faite pour rembourser, non pour investir. C'est une dette toxique ! Comment un Français qui chaque mois compte Comment un Français qui chaque mois compte et limite ses dépenses peut-il comprendre ? Comment peut-il comprendre que l'argent n'a pas de valeur, alors qu'il s'efforce tous les jours de faire attention ? Monsieur le ministre, je ne supporte plus l'utilisation que vous faites de l'argent public, de l'argent qui ne vous appartient pas ! Je ne supporte plus le fait que vous soyez incapable de réduire les dépenses et de diminuer les normes et les contraintes administratives qui engendrent l'augmentation- contrairement à vos prévisions Les dépenses ne sont pas maîtrisées et le service public ne cesse de se dégrader. Les Français se plaignent à juste titre de la lenteur et de l'inefficacité de la justice, les forces de l'ordre s'épuisent et se découragent, l'immigration augmente sans aucun contrôle.

d'intérêts serait bientôt insupportable, dépassant le budget de la défense, pourtant deuxième budget de l'État. La Cour des comptes, le Haut Conseil des finances publiques et le Sénat vous mettent en garde, mais vous n'écoutez pas.

du modèle de financement des collectivités doivent désormais primer la réforme fiscale des collectivités en tant que telle. Je passe évidemment, bien que ce sujet demeure fondamental, sur la réforme des critères d'attribution de la DGF et sa singulière complexité. Mais nous aurons ce débat ; l'examen des articles portant prélèvement sur recettes au profit des collectivités en sera certainement l'occasion. Un commentaire, enfin, sur la méthode et sur la trajectoire.

Que des injonctions contradictoires trouvent à s'exprimer entre les interventions de représentants de différents groupes, c'est assez logique. J'entends parfois aussi des injonctions contradictoires au sein des mêmes groupes, et j'ai souvent constaté que les mêmes qui, en discussion générale,

Madame la présidente, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, nous passons désormais à l'examen de l'article 18 du projet de loi de finances pour 2022, qui évalue à 26,4 milliards d'euros le montant du prélèvement sur recettes versé par la France au profit de l'Union européenne- somme relativement stable par rapport à la prévision actualisée pour 2021. cette relative stabilisation ne saurait refléter l'amorçage d'un plafonnement ni d'un ralentissement de la contribution française. En effet, le montant annuel moyen de ce prélèvement devrait s'élever à 27,6 milliards d'euros pour la période 2021-2027, soit une hausse de 7,5 milliards d'euros par rapport au montant moyen acquitté pour la période 2014-2020. Cela étant dit, il convient de rappeler que la France reste l'un des principaux bénéficiaires en volume des dépenses de l'Union européenne, en deuxième place derrière la Pologne. Ainsi, en 2020, les dépenses réalisées en France se sont élevées à 15,8 milliards d'euros, soit près de 11 % des dépenses totales de l'Union, en hausse de 5,4 % par rapport à l'année précédente. Au-delà de la question du montant de la contribution de la France pour 2022, les auditions que j'ai menées m'ont permis d'identifier trois défis auxquels le budget européen devra répondre dans les prochaines années. Premièrement, alors qu'un nouveau cadre financier pluriannuel vient de s'ouvrir, il faut veiller à ne pas manquer le coche du démarrage de cette nouvelle programmation, afin de mobiliser de façon efficace les fonds européens, sujet auquel le Sénat est attaché. Or l'allongement du délai entre l'engagement des dépenses et leur paiement se traduit par une hausse du reste à liquider, qui s'élève à 300 milliards d'euros environ à la fin de l'année 2020. Certes, la constitution d'un reste à liquider est un phénomène normal, mais son excès témoigne d'une difficile concrétisation des dépenses européennes sur le terrain. alors que la mission d'information du Sénat sur ce sujet a rendu ses conclusions voilà maintenant deux ans, quelles mesures concrètes le Gouvernement a-t-il prises pour accélérer la mobilisation des fonds européens dans les territoires ? Deuxièmement, la présentation des propositions de la Commission européenne pour l'introduction de nouvelles ressources propres a été repoussée à une date ultérieure. l'introduction de nouvelles ressources nous a été présentée comme la voie permettant de financer le remboursement du plan de relance européen, mis en oeuvre grâce à une nouvelle capacité d'endettement commune.

rien qu'au titre du remboursement du plan de relance. Monsieur le secrétaire d'État, face à l'urgence de ce dossier, pouvez-vous nous donner des perspectives quant au calendrier des propositions qui doivent être émises par la Commission européenne ? Troisièmement, la Commission européenne a présenté en juillet le paquet Climat. Il y est notamment proposé qu'une partie des recettes du système d'échange de quotas d'émission alimente un fonds social pour le climat, destiné à alléger la facture énergétique des ménages et des entreprises. Par conséquent, deux objectifs seraient désormais attribués à cette même ressource rembourser le plan de relance européen et financer le fonds social pour le climat. Monsieur le secrétaire d'État- et ce sera ma dernière question -, alors que les nouvelles ressources propres ne sont pas encore arrêtées, faut-il déjà s'inquiéter d'un risque de dévoiement de ces recettes au détriment du remboursement du plan de relance ? Enfin, l'examen du montant du prélèvement sur recettes m'a donné l'occasion, en commission, de faire un point sur la mise en oeuvre du plan de relance européen, au titre duquel la France a déjà bénéficié du versement du préfinancement, pour un montant de 5 milliards d'euros environ.

et de résilience des États membres. Je souhaiterais néanmoins relayer un point de vigilance sur le recours aux crédits de la facilité pour la reprise et la résilience en France. En effet, ces crédits peuvent financer des mesures qui sont également éligibles aux fonds de la politique de cohésion. Or une même dépense ne peut être financée par plusieurs fonds. Il faut donc mettre en place un système d'aiguillage, ou de priorité, pour flécher les financements. L'enjeu budgétaire est de taille. Si nous voulons utiliser pleinement tous les crédits alloués à la France, les financements doivent être bien fléchés. À l'heure actuelle, une démarche pragmatique semble être privilégiée, mais il nous reviendra de suivre attentivement cette mise en oeuvre. En conclusion, mes chers collègues, je recommande, au nom de la commission des finances, l'adoption sans modification de l'article 18 du projet de loi de finances pour 2022. La parole

monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, je veux tout d'abord excuser le président Jean-François Rapin et remercier notre collègue Jean-Marie Mizzon pour son analyse et pour la clarté de ses propos. Il nous a indiqué que la contribution de la France au budget européen était stabilisée.

à rembourser l'emprunt contracté à l'occasion du lancement du plan de relance européen. Il existe, bien sûr, une échappatoire à cette perspective : la mise en place de nouvelles ressources propres.

C'est un fait, et la commission des affaires européennes entend s'y intéresser tout particulièrement l'an prochain, dans le cadre de la présidence française du Conseil de l'Union européenne. Monsieur le secrétaire d'État, peut-être pouvez-vous nous apporter des précisions sur ce point ? Mardi dernier, le ministre Jean-Yves Le Drian a évoqué trois mots d'ordre pour qualifier les ambitions de la future présidence française : relance, puissance, appartenance. Acceptons-en l'augure, mais je veux ici affirmer que, si les attentes du Sénat sont grandes, ses doutes n'en sont pas moins grands quant à la capacité de la France de tirer le meilleur parti de cette présidence, en raison du calendrier électoral. Pour ce qui est de la relance, nous pouvons dire que nous l'avons financée à crédit, tant au niveau national qu'au niveau européen. La puissance, elle, reste largement à construire et exige une véritable volonté politique.

Il faut parvenir à traduire en actes l'affirmation de l'autonomie stratégique de l'Union, c'est-à-dire donner corps et sens au projet européen, en pensant d'abord à nos concitoyens ; à défaut, ces derniers s'en détourneront. Nous avons tous les jours des exemples indiquant que ce risque est réel. Cela vaut pour le Pacte vert et la transition écologique comme pour les enjeux migratoires ou la défense, pour ne citer que quelques exemples. La commission des affaires européennes et l'ensemble des commissions permanentes, dont je salue la mobilisation, entendent utiliser pleinement le volet parlementaire de la présidence française pour veiller à la défense des intérêts de la France et faire en sorte que les attentes des citoyens européens soient pleinement prises en compte par les institutions européennes. La parole

cours du débat que le Sénat y a consacré mardi, certains de mes collègues ont souligné la peu idéale concordance entre cet événement et la prochaine élection présidentielle. Voyons les choses autrement reprise économique, pandémie, migration, transition écologique, sécurité internationale, ces sujets n'ont pas de frontières et, pour la plupart, appellent une réponse à l'échelle du continent européen- c'est une évidence, en tout cas aux yeux du RDSE, profondément attaché, chacun le sait, à la construction communautaire. La campagne présidentielle devra donc être l'occasion de rappeler à nos concitoyens, et surtout aux plus eurosceptiques d'entre eux, cette interdépendance entre le destin de la France et celui de l'Europe. Regardons la reprise économique, dont la France profite particulièrement une telle dynamique aurait-elle été possible sans le plan de relance et l'effort coordonné de mutualisation des dettes ? La stratégie vaccinale européenne mérite également d'être évoquée. L'approche collective a permis de sécuriser l'approvisionnement en doses sur notre continent. Ainsi, une grande majorité des États membres de l'Union européenne figurent parmi les pays les mieux vaccinés au monde. Cela dit, je n'oublie bien sûr pas les terrains sur lesquels des efforts restent à faire en faveur d'une approche plus coopérative.

combien piétine le paquet Migration et asile. Pourtant, les défis sont immenses, entre le désespoir qui pousse les migrants à quitter leur pays et l'instrumentalisation honteuse qui est faite de ce drame par certains États, hier le Maroc, aujourd'hui la Biélorussie. Mes chers collègues, pour amplifier ces politiques, comme chaque année, notre pays doit s'acquitter de sa quote-part au budget de l'Union européenne. Nos collègues rapporteurs ont rappelé les chiffres : en 2022, le prélèvement sur les recettes de l'État au au profit de l'Union s'élèverait à 26,4 milliards d'euros, soit 800 millions d'euros de moins qu'en loi de finances initiale pour 2021. Au regard de cette somme, la question du juste retour est dans les esprits

Quoi qu'il en soit, il faudra en finir un jour avec les rabais, lesquels vont à l'encontre du principe de solidarité qui est au fondement du projet européen. Le remboursement de l'emprunt pourrait être l'occasion d'approfondir le financement du budget de l'Union européenne. Mon groupe partage les orientations qui sont sur la table depuis l'accord du Conseil européen de juillet 2020 : taxe numérique, produit du système d'échange de quotas d'émission ou encore mécanisme d'ajustement carbone aux frontières.

Madame la présidente, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, chaque année, nous débattons de la contribution de la France au budget de l'Union européenne. Ce moment, sans doute trop court, nous permet aussi d'aborder l'état de l'Union.

ainsi gelé l'application des règles de la discipline budgétaire, notamment les fameux seuils de 3 % du PIB pour le déficit public et de 60 % du PIB pour la dette publique, et assoupli les critères encadrant l'octroi d'aides d'État.

Toutes ces décisions ont eu un fort impact sur le budget de l'Union européenne, contribuant à limiter l'augmentation attendue de la participation française à ce budget. Cette pandémie a également révélé la nécessité d'un changement de politique de grande envergure. Nous n'avons plus le choix : nous devons désormais nous prémunir contre les crises à venir protéger les plus vulnérables. Il nous faudra atténuer, voire résoudre, les crises, qu'elles soient sociales, économiques, écologiques ou démocratiques, et résorber les inégalités qui fragilisent nos sociétés. Il est aujourd'hui urgent de redéfinir un cadre budgétaire et monétaire européen durable et de rebâtir nos politiques à la hauteur des enjeux qui sont devant nous.

Aujourd'hui, l'Union européenne doit trouver d'autres financements que la contribution des États membres ou l'emprunt sur les marchés financiers. La Commission européenne a d'ailleurs proposé, le 14 juillet dernier, l'instauration d'un mécanisme d'ajustement carbone aux frontières et le renforcement du système d'échange de quotas d'émission. Ces ressources propres favorables à l'environnement prolongeraient la démarche et l'esprit qui ont présidé à la mise en place de la taxe sur les déchets

qui permettrait à la France de récupérer un montant de l'ordre de 25 milliards d'euros de recettes, accroissant de manière significative notre capacité budgétaire. Cet accord international condamne-t-il toute possibilité d'atteindre rapidement

afin de renforcer la transparence et ainsi de mettre un terme à ces pratiques fiscales dommageables. Chaque année, les gouvernements européens perdent plus de 1 000 milliards d'euros de recettes en raison des pratiques de fraude et d'évasion fiscales de la part d'entreprises et de

Rappelons que le 1 % des individus les plus riches détient 20 % à 25 % de la richesse totale en France, en Allemagne, en Espagne ou encore en Scandinavie. Dès lors, pourquoi ne pas taxer aujourd'hui leur richesse nette et leur capital de manière de manière progressive, à l'échelle de l'Union européenne ? Ces recettes nouvelles pourraient être consacrées au remboursement des euro-obligations émises lors de la crise sanitaire, à la constitution d'un fonds commun de sauvetage ou à la transition environnementale, qui est notre horizon. Cet impôt concernerait l'accumulation passée ; les rendements de l'investissement actuel et de l'innovation ne seraient donc pas affectés. Il ne représenterait donc un frein ni à l'investissement ni à la reprise. Ce 1 % des Européens aiderait ainsi les 99 % restants ! Des voies s'offrent à nous à nous de les saisir. Aujourd'hui, le groupe socialiste votera la contribution proposée dans ce budget pour 2022, qui est indispensable à la solidarité européenne, tout en appelant également à la construction d'une Europe forte, unie, fondée sur l'équité sociale et engagée dans les transitions, la

l'an dernier, j'avais ouvert mon propos en évoquant la violence de la crise que nous traversions et les blocages qui subsistaient dans les négociations du nouveau cadre financier pluriannuel 2021-2027. Force est de constater que la crise est loin d'être terminée et que d'autres blocages, héritiers de situations latentes, se sont créés au sein de l'Union européenne. Ce qui n'a pas changé non plus, c'est le montant de la contribution annuelle française au budget de l'Union, qui dépasse à nouveau les 26 milliards d'euros. L'Union européenne fait énormément pour nos territoires et pour chacun d'entre nous au quotidien, quotidien, grâce à des financements importants ; de surcroît, jour après jour, nous lui demandons d'agir toujours davantage. Nous sommes d'ailleurs, depuis des années, l'un des principaux bénéficiaires des dépenses de l'Union. C'est particulièrement le cas pour la politique agricole commune (PAC), qui tient une place prépondérante dans les fonds européens que nous recevons et contribue à la force de notre agriculture et à notre souveraineté alimentaire.

Dans cet hémicycle, en février dernier, nous avons ratifié la décision « ressources propres » ; elle prévoit notamment un calendrier. Certaines délibérations devront se tenir durant la présidence française du Conseil de l'Union européenne. Nous comptons sur le Gouvernement, monsieur le secrétaire d'État, pour mener des discussions efficaces et faire émerger des solutions pérennes. L'enjeu est trop important pour être remis à plus tard. 2028 sera la première du remboursement de notre dette commune ; autant dire que c'est demain. Surtout, 2028 marquera le début d'un nouveau cadre financier pluriannuel, qu'il faudra négocier, qui se traduira par de nouvelles contributions annuelles françaises. de l'argent de la prochaine génération, qui fera face à de nombreux défis. Alors que notre jeunesse nous exhorte à prendre des décisions dans d'autres domaines, notamment sur le climat, avec la COP26 qui s'est achevée, nous devons prendre nos responsabilités sur les volets économique et financier. Là aussi, il y a urgence : des ressources propres solides sont nécessaires.

L'Union européenne n'est pas une option ; c'est un levier indispensable pour faire face aux défis actuels. La parole le groupe Les Républicains

Le prélèvement sur recettes est donc un geste financier fort, un engagement politique sans équivoque. En responsabilité, puisqu'il s'agit tant de satisfaire à une obligation internationale de la France que de permettre le fonctionnement de l'Union européenne, le groupe Les Républicains y souscrira et votera donc l'article 18 qui nous est soumis aujourd'hui. Le traditionnel débat sur le prélèvement sur recettes intervient toutefois cette année dans un contexte très particulier, marqué par le lancement effectif du plan de relance européen approuvé en juillet 2020. Cet accord avait fait tomber l'un des grands tabous de la construction européenne en autorisant pour la première fois un endettement commun à grande échelle. Une condition, toutefois, clairement explicitée par les chefs d'État et de gouvernement : le plan de relance, donc le pouvoir d'emprunt sur les marchés conféré à la Commission, doit demeurer « une réponse exceptionnelle à des circonstances temporaires Or le Gouvernement prend désormais des distances de plus en plus marquées avec cette clause, dont l'objectif était d'affirmer que l'Europe ne s'engagerait pas à bas bruit sur la voie du fédéralisme budgétaire à la faveur de sa réponse aux conséquences de la crise sanitaire. Alors même que les premiers décaissements n'avaient pas encore été effectués, Bruno Le Maire déclarait ainsi au mois de juillet : « nous proposons que l'émission de dette en commun réalisée pour financer le plan de relance devienne un système permanent de financement européen. En échange, chaque État membre accepterait d'être plus responsable en matière de dépense publique ». En premier lieu, permettez-moi de souligner que l'exigence de sérieux budgétaire figure déjà depuis de nombreuses années au coeur du pacte de stabilité et de croissance et du pacte budgétaire. Par ailleurs, je crains que l'exemple de ce projet de loi de finances, qui ne cesse d'évoluer au rythme effréné des promesses présidentielles, n'incite guère nos partenaires à se ranger aux propositions françaises. Quoi qu'il en soit, monsieur le secrétaire d'État, pouvez-vous nous confirmer que la position défendue à Bruxelles par le Gouvernement est bien celle d'une pérennisation du système d'endettement commun ? Dans l'affirmative, pouvez-vous nous donner un ordre de grandeur des volumes financiers Autre élément central de l'accord sur le plan de relance, la question des ressources propres est, comme on pouvait s'y attendre, loin d'être réglée. À vrai dire, au-delà de l'accord de principe donné par le Conseil européen, le débat de fond n'a même pas véritablement débuté. En effet, la feuille de route contenue dans l'accord interinstitutionnel de décembre 2020 prévoyait que la Commission ferait une première série de propositions au plus tard en juin 2021, pour une entrée en vigueur des nouvelles ressources propres au 1 janvier 2023. Or ce calendrier est déjà dépassé. Le projet de ressource assise sur une redevance numérique, dont une première version avait été présentée en 2018, puis abandonnée faute de consensus, a ainsi été mis en pause à la suite de l'accord conclu à l'OCDE sur la fiscalité des grandes entreprises. Quant au mécanisme d'ajustement carbone aux frontières et à la révision du système d'échange de quotas d'émission, ils figurent bien dans le paquet climatique « Ajustement à l'objectif 55 » présenté le 14 juillet par la Commission. a toutefois choisi de n'établir, à ce stade, aucun lien entre ces instruments et la décision sur les ressources propres de l'Union, au grand dam, d'ailleurs, du commissaire au budget et à l'administration, Johannes Hahn, qui n'a pas hésité à faire part de son mécontentement.

Les discussions à venir seront donc ardues et rien ne garantit qu'elles aboutissent. Le parcours chaotique de la taxe sur les transactions financières et de l'assiette commune consolidée de l'impôt sur les sociétés nous incite en effet à la prudence engluées dans des débats sans fin depuis des années, celles-ci sont pourtant censées abonder le budget européen dès le 1 janvier 2026. L'enjeu n'est pas mince, puisque la charge du remboursement du plan de relance sera de plus de 15 milliards d'euros par an

de plus de 2,5 milliards d'euros par an, soit une hausse de près de 10 % par rapport au prélèvement sur recettes que nous examinons aujourd'hui. Dans ces conditions, le plan européen allouerait certes 40 milliards d'euros de subventions à notre pays, mais il lui demanderait, en contrepartie, de rembourser plus de 70 milliards d'euros. Un bien mauvais calcul, en somme, pour la France, qui sera en outre le principal contributeur au financement des rabais- 53 milliards d'euros sur sept ans -que les États frugaux ont réussi à conserver, et dont ils ont même obtenu l'augmentation, en échange de leur soutien à la relance européenne. Je conclurai mon propos en évoquant brièvement l'après-plan de relance et la consultation lancée récemment par la Commission européenne sur la révision des règles du pacte de stabilité et de croissance. La clause dérogatoire générale activée en mars 2020, qui permet aux États membres de s'extraire des règles en matière budgétaire et d'aides d'État, a été prolongée jusqu'à la fin Cette orientation budgétaire expansionniste ne pourra toutefois durer éternellement et les finances publiques nationales devront, tôt ou tard, retrouver une trajectoire soutenable, en particulier dans les pays très lourdement endettés, comme la France. Il importe de préparer l'avenir en pensant aux générations futures qui auront à rembourser notre dette sans forcément en avoir la capacité. Il importe également que la France, qui s'apprête, en janvier prochain, à prendre la présidence du Conseil de l'Union européenne, soit exemplaire en matière de gestion de ses finances publiques. Le débat sur la manière dont le pacte de stabilité et de croissance devra trouver à s'appliquer de nouveau fera, à n'en pas douter, l'objet de très nombreuses propositions. Il ne faudra toutefois pas perdre de vue certains fondamentaux essentiels pour préserver tant la solidité que la compétitivité de la zone euro. Si le cadre révisé pourra éventuellement faire preuve de davantage de souplesse et de réactivité, il n'en devra pas moins rester suffisamment strict pour assurer, dans chaque État membre, le retour à des niveaux soutenables de dépense et de dette.

en déplafonnant le budget européen du fameux 1 % du PIB, en décidant d'un emprunt commun pour la relance et en lançant la démarche pour l'introduction de nouvelles ressources propres. C'est bien une véritable capacité budgétaire européenne, j'y insiste, qui a été rendue possible. le cadre financier pluriannuel dans lequel nous sommes engagés est d'une ampleur nettement différente du précédent. Le choix commun de consacrer directement près du tiers de nos moyens au climat sera déterminant pour tenir l'objectif d'une réduction

disons-le : Glasgow, quel gâchis ! Quelle incapacité de l'Europe à se montrer unie, résolue et entraînante ! L'Europe aura surtout étalé publiquement ses divisions sur le caractère positif ou négatif des investissements gaziers, pétroliers et nucléaires, la France, qui arrange son alliance entre tenants du nucléaire et tenants des hydrocarbures, et cinq États, dont l'Allemagne, qui la critiquent vertement. On est loin de la cohésion la cohésion européenne des COP précédentes ! Il va pourtant bien falloir retrouver un tel esprit de cohésion si l'Union veut affronter les trois défis majeurs que sa résolution budgétaire nouvelle de juillet 2020 le déploiement effectif de la relance sans que se dénaturent les orientations majeures, climat, énergie, santé, économie durable et résiliente, transition numérique, justice sociale, ni que se dévaluent les valeurs qui cimentent l'Union, lesquelles

d'emprunter pour investir dans les transitions d'avenir et la neutralité carbone. La clause dérogatoire générale du pacte de stabilité et de croissance devrait être levée dans un an contre-productif de rétablir les verrous d'hier. La présidence française est attendue sur ce point et l'approche qu'adoptera la future coalition outre-Rhin sera déterminante. Enfin, troisième défi : la création de nouvelles ressources propres. L'emprunt commun nous y oblige, à moins d'augmenter les contributions des États ou de ratiboiser les politiques de l'Union. L'accord pour le déploiement des ressources propres

patine, dans le contexte nouveau de l'accord fiscal international, les perspectives restant confuses. Ce qui est bien moins confus, après la publication des, c'est la réalité de l'évasion fiscale : voilà, là aussi, des ressources à collecter avec détermination.

Madame la présidente, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, il aura fallu, nous dit-on, une pandémie mondiale pour estomper les égoïsmes nationaux incarnés par les pays dits « frugaux L'accord faussement historique du plan de relance européen, entre autres cérémonies d'autosatisfaction, empêche de prendre la mesure de la crise qui traverse l'Europe. Opposant les plus frugaux aux moins frugaux, le débat se mène entre frugaux

Les frugaux donnent le la, la France semble subir. La contribution française pour l'année 2022 s'élève à 26,4 milliards d'euros, soit un quart de plus qu'en 2014, à périmètre constant. Les États membres se trouvent traversés par des désaccords sur les orientations politiques et sur les moyens qu'ils sont prêts à concéder. Ces divergences engendrent confusions, renonciations et tentatives de justifications J'en

lenteur dans le versement des crédits pourrait s'avérer extrêmement dommageable dans un contexte de relance. Bénéficierons-nous de ces crédits, ou bien devrons-nous y renoncer ? Tablons-nous

Le plan de relance français se déroule sans ces crédits, sans que cela semble poser le moindre problème de financement. Nous maintenons cette appréciation. Troisièmement, le rendez-vous est fixé à 2028 pour le début du remboursement.

par manque de courage politique et à cause de la marginalisation de la France sur la scène européenne, malgré une mise en scène rondement menée. La présidence française du Conseil de l'Union européenne, dont on ne sait pas grand-chose à l'heure qu'il est, sera elle aussi entravée par les frugaux tant que le Président ne résoudra pas un paradoxe majeur : il lui faut porter la conquête sur de nouvelles ressources européennes, alors même qu'il se refuse à entendre parler de nouvelles recettes

Ce prélèvement opéré sur les recettes du budget de l'État, dont le montant représente actuellement 26,4 milliards d'euros, auxquels il faut ajouter les droits de douane, constitue l'élément essentiel de la participation française au budget européen. Avant toute chose, je tiens à remercier Jean-Marie Mizzon, notre rapporteur spécial, pour la qualité du travail qu'il a accompli. Le budget de l'Union européenne pour l'année 2022 s'élève à 169,4 milliards d'euros, hors paiements au titre de la réserve d'ajustement au Brexit. de paiement augmentent de 2 % par rapport à 2021, en raison notamment d'une montée en puissance de nouveaux programmes d'investissement, de santé et d'action extérieure. Nous pouvons nous féliciter que les priorités fixées au sein du cadre financier pluriannuel 2021-2027 soient respectées.

des crédits alloués au programme Erasmus+, qui demeure l'un des dispositifs les plus connus et appréciés de nos concitoyens, notamment des plus jeunes d'entre eux. Pour en revenir à la participation de la France au budget européen, celle-ci se caractérise par une relative stabilité, justifiée par la contribution accrue de Londres au titre de ses obligations financières post-Brexit et par l'accroissement des droits de douane, qui est directement lié au rebond économique de notre pays. Ces données ne doivent pas occulter trois facteurs politiques et économiques favorisant la hausse systématique,

mais aussi les difficultés à analyser l'impact de la nouvelle taxe plastique en 2021, ainsi que les différents rabais, auxquels il a déjà été fait allusion, négociés par cinq États membres- l'Allemagne, les Pays-Bas, la Suède, l'Autriche et le Danemark. Ce dernier point doit évidemment faire l'objet d'une attention À une époque où l'idée de solidarité européenne est brandie à tout-va, ces dérogations budgétaires tendent toujours à favoriser la défiance, voire la mésentente, entre États membres. Aussi le budget pour 2022 s'accompagne-t-il d'un lot de défis à relever. Pour commencer, comme cela a été réaffirmé à plusieurs reprises, y compris en commission des finances le 27 octobre dernier, l'instauration de nouvelles ressources propres est un impératif absolu. Qu'il s'agisse d'une redevance numérique, d'un mécanisme d'ajustement carbone aux frontières ou d'une taxe sur les transactions financières, les négociations doivent reprendre et aboutir. Les pistes de réforme étudiées à l'échelle de l'OCDE ne sont pas incompatibles avec des travaux menés au niveau européen. Ce point est d'autant plus crucial que les produits des nouvelles ressources propres serviront à financer le plan de relance européen. Si des avancées en matière de

Par ailleurs, l'annonce en juillet dernier d'un objectif de réduction de 55 % des émissions de gaz à effet de serre de l'Union européenne d'ici à 2030 doit se traduire par l'affectation d'une partie des nouvelles ressources propres à un fonds social pour le climat.

je veux également attirer votre attention sur la hausse structurelle du reste à liquider, symptôme d'un allongement du délai entre l'engagement des dépenses et leur paiement.

Les démarches doivent être simplifiées afin que les crédits européens soient rapidement et efficacement alloués. Tous ces défis devront être relevés à l'occasion de la future présidence française de l'Union européenne, dont nous attendons encore la feuille de route précise,

Comme le disait Jacques Delors après la crise des de 2008, « après les pompiers, l'Union européenne attend les architectes ». Telle sera la mission de la présidence française. Nous attendons donc, monsieur le secrétaire d'État, des réponses qui redonnent du souffle et des initiatives qui « reboostent » l'envie d'Europe de nos concitoyens ; plus encore, nous attendons la vision d'une Europe qui protège

je crois pouvoir dire que la solidarité budgétaire en Europe a connu des avancées importantes. Je vais en dire un mot en répondant à quelques-uns des points qui ont été soulevés dans la discussion. D'abord, cette solidarité européenne a été actée

Ce débat est essentiel, car il fait partie, avec le plan de relance, de la stratégie de croissance et d'investissement de l'Union européenne. L'application des règles- cela a été rappelé -est suspendue jusqu'à la fin de l'année 2022 ; cela signifie que nous devons anticiper le retour à la normale

Nous pouvons sans doute encore améliorer les choses, mais je tiens à préciser que nous avons souhaité- j'ai souhaité personnellement -une association transpartisane à la préparation de cette présidence. À trois reprises déjà s'est réuni un comité transpartisan, où siège un représentant de chaque groupe de votre assemblée comme de l'Assemblée nationale et du Parlement européen.

J'informe le Sénat que la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure est parvenue à l'adoption d'un texte commun.